La séance est reprise nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Dans la discussion des articles nous sommes parvenus à l'article 8. Et sur cet article que nous avons une demande de parole de madame Gisèle Jourda. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le président, mes chers collègues, c'est à la Lina 15 de cet article 8 que nous avons fait adopter en commission des amendements tendant à préciser le bilan annuel relatif à la mise en oeuvre des objectifs concernant les réserves. Il devra désormais rendre compte du développement de l'attractivité de la réserve pour les salariés et les étudiants et dresser un état d'avancement des conventions de partenariat signé entre le ministère de la Défense et d'une part les entreprises d'autre part, les établissements d'enseignement supérieur. En janvier 2020, ce sont près de 850 employeurs privés ou publics qui ont signé une convention de soutien à la politique de réserve militaire. Si l'on considère qu'il existe plus de 3 millions d'entreprises en France. La marge de manoeuvre Paris réel à la vérité. Le changement impulsé dans ce domaine semble avant tout une affaire de mentalité et le travail à mener est celui d'une sensibilisation accrue aux enjeux de la réserve militaire il aime. De faire comprendre aux employeurs que l'activité au sein de la réserve opérationnelle ouvre un processus triplement gagnant pour les armées pour le réserviste mais aussi pour les employeurs, compte tenu de l'enrichissement des qualités compétences ce savoir-faire et acquis les des réservistes que qui peuvent directement être bénéfique à l'entreprise cette valeur immatérielle des réservistes méritant d'être mieux reconnues. Nous avions préconisé également de dévolu. L'acteur activité de la réserve envers les étudiants en sensibilisant les chefs d'établissement à la dimension formatrice et au potentiel d'intégration professionnelle que comporte pour un étudiant sa participation à la réserve. Monsieur le Ministre, à l'heure actuelle, combien d'établissements ont signé une telle convention, nous sommes nombreux dans cet hémicycle, a souhaité une intensification des démarches visant à étreindre ses partenariats entre le monde de la défense et de l'entreprise. Merci beaucoup madame Jourda. La parole est à monsieur tu es mal pour l'amendement 70. Ou l'amendement porte-avions quoi comme vous voulez, en fait l'idée c'est que nous estimons que pour faire notre nous remplir nos missions. Il y a il y a il y a un sujet d'informations de connaissances et c'est vrai que dans les débats que nous avons eu en préparation de la LPM.

Si Monsieur es mal monsieur le rapporteur. Monsieur le président. Mais merci madame la présidente. L'objectif de cet amendement et et tout à fait raisonnable, et je pense que c'est bien évidemment comme on l'a dit à plusieurs reprises déjà au cours de cet après-midi c'est le rôle du sénat de faire en sorte de s'informer et d'obtenir les informations sur les coûts complets des programmes. Bien évidemment, je pense que nous pouvons aussi utiliser les pouvoirs propres de la déco de notre commission permanente et singulièrement les Hauts-de-Seine. Selon les investigations sur pièces et sur place et en l'occurrence et tout à fait normal que sur un équipement aussi important que le futur porte-avions on puisse avoir une estimation du coup j'ai je sais que ça avait écrit ça avait créé au sein de la commission un certain émoi, ne pas recevoir des plus hautes autorités une réponse concrète mais enfin bon je pense que cet amendement d'appel l'appel a été entendu et. Parce qu'il est possible de de de retirer. De retirer ce en demandant, bien évidemment au ministre de nous donner tous les éléments pour satisfaire la curiosité de du président est mal. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre avait du gouvernement. Oui merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur optimal ah amendement d'appel de fait. il y a déjà beaucoup de choses, on n'est pas appelé rap ça c'est quand même un des éléments qui m'avait frappé lors de la discussion budgétaire. Lors de la défense des crédits pour 2023 l'Automne dernier c'est que bon nombre de questions des parlementaires, Assemblée, Sénat. Figurer en fait dans les documents qui était obligatoire de par la LOLF pas tout le temps mais je, je le précise quand même. Et en fait ce que j'ai indiqué d'ailleurs ou de président et bon et où c'est que à un moment donné, je pense que ça vaut le coup aussi de de de bien. Tracer les informations dont vous avez vraiment besoin la programmation militaire le Champ est infinie. Donc le Champ de la documentation l'est tout autant qu'on fait le, l'engagement que j'ai pris devant le président Gontard tout à l'heure sur les questions. Des carburants enfin bon donc il y a des sujets spécifiques. Typiquement, on y reviendra tout à l'heure sur le porte-avions sur le la la prolongation du Charles-de-Gaulle. Une réponse adéquat peut être par un sous-, un moment d'ailleurs, si vous le souhaitez, on pourra évidemment travailler ça donc je pense que ce que vous que vous avez décidé en commission, c'est-à-dire le rapport annuel sur l'exécution de la LPM est un bon moyen de sérier déjà les questions que vous voulez adressé à l'exécutif ou le cas échéant aux états majors. Donc en tout cas moi je suis disponible. Je l'ai dit tout à l'heure à la tribune typiquement sur la disponibilité du matériel, c'est une avancée il y a des sujets qui sont classifiés. On le comprend très bien. Bref. autre point j'essaierai pour la discussion budgétaire, une innovation, j'en ai parlé à au président Cambon. Quand on dit rapport, tout d'un coup pour Balard pour les états majors, c'est beaucoup de choses parfois une note flash toute simple. Comme le disait que j'ai encore bon, un bon tableau peut valoir. Voilà donc on peut aussi avoir une réflexion collective par consensus entre les groupes en se disant est-ce qu'on fait pas aussi évoluer la forme de ce qui est fourni. Parce que de l'autre côté de la barrière, je vois aussi des équipes qui travaillent beaucoup à produire des documents et donc je pense qu'on peut peut-être trouver un modus Vivendi font forme qui permet d'être efficace. Voilà en tout cas je pense que c'est un bon débat pour l'avenir. Il y a les sujets le le FICC 1er sujet les sujets propres aux mines, armes à la programmation militaire et je pense qu'en fonction aussi moi je vois bien entre Assemblée Sénat vous ne vous intéressez pas la même chose donc de fait, ça fait deux exercices qui sont différents. C'est ça qui faisait de cadrer. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur Il est retiré. Je vous remercie. L'amendement 70 s'est retiré, amendement 150, madame Gréaume. Merci madame la présidente. L'article 8 prévoit la remise par le gouvernement d'un rapport annuel sur le bilan d'exécution de la LPM adressée aux commissions permanentes des deux chambres. Je crois que nombre de nos collègues dans tous les groupes partagent l'exigence d'une information la plus complète du Parlement. C'est une condition indispensable pour nous permettent de faire notre travail, c'est-à-dire de contrôler l'action du gouvernement et c'est ce qu'on a discuté déjà. Tout à l'heure. Trop souvent, nous recevons des données au compte-goutte de manière partielle. J'ajoute que le motif, secret défense et de plus en plus opposés à nos demandes de précisions. Aussi, afin de préciser encore les attendus du rapport. Nous proposons d'y inclure un bilan d'exécution des opérations extérieures, suivi d'un vote à bilan spécifiques concernant la protection de la souveraineté des territoires ultramarins et enfin un bilan des opérations des des pollutions relatives aux déchets nucléaires en Polynésie française. Il nous semble en effet important de permettent le débat parlementaire sur les OPEX, dont le nombre et le coût ont fortement augmenté, ainsi que sur les enjeux relatifs aux territoires ultramarins où beaucoup d'attentes s'exprime, y compris à l'occasion de cette LPM merci. Merci madame. Monsieur le rapporteur. Avis de la commission. Merci madame la présidente. La Commission pense qu'il n'est pas utile de multiplier les sujets sans lien Direct et immédiat avec l'exécution de la loi de programmation militaire sur les points abordés par cet amendement. Je rappelle que le contrôle parlementaire des OPEX et est organisée et fixé par l'article 35 de la Constitution et que rien ne nous empêche, ce que nous avons encore fait récemment d'organiser des débats. La présence de la France en Afrique avait un volet très important sur ce sujet. De la même manière sur le déroulement des programmes. Et le renforcement des moyens basés dans les outre-mer le bilan d'exécution de la LPM va nous permet de suivre ce déroulement enfin les conséquences des essais nucléaires français dans le Pacifique. C'est une question importante. Nous ne négligeons pas l'impact et dont qui nous préoccupe, bien sûr, mais cette disposition n'a pas sa place à l'article 8 de la LPM, donc c'est un avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente, madame la sénatrice. Sur les 3 aspects OPEX, pour moi c'est déjà couverts par les dispositions de l'article 4 objectivement. Plus les auditions que vous avez avec les différents jeux d'État-Major votre serviteur et cetera sur souveraineté des territoires ultramarins objectivement l'article 8 permet de le, de le couvrir. Si vous estimez qu'il fallait que je prenne un engagement supplémentaire en fonction de 2 points précis ce que vous attendez sur l'outre-mer évidemment j'y suis pas opposé. Il y a pas de secret défense pour le coup en la matière, c'est moins que l'on puisse dire et sur les dépollution nucléaire. Dans le bilan environnementaux tu es qui sont précisés. L'article 8 je me suis engagé. Vis-à-vis des députés de Polynésie française, à l'Assemblée nationale à ce que dans ses rapports de l'article 8, le volet des pulsions soit. Comment dire, intégrait on a eu un peu d'échange

Madame Gréaume. Il est retiré le 150 et donc retiré et je mets aux voix l'article 8. Qui pour. Qui compte. Qui s'abstient. Il était adopté. Article 9, nous avons l'amendement 243 du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui mais la présente, il est purement rédactionnel parce que le référentiel physico-financier de programmation militaire on on y met ce qu'on a envie je pense que l'intention du législateur, c'était des chroniques de commandes et de livraisons des principaux. En tout cas physique ou financier programmation militaire si ça reste en l'état, ce ne sera pas un drame, mais ça sera tellement flou que le gouvernement à l'avenir parce que ce sera pas forcément toujours votre serviteur pour émettre ce qu'il aura envie. Donc je pense que l'amendement du gouvernement permet au final d'être un peu plus sévère encore que que le Parlement avait prévenu

et puis au titre du bilan annuel prévu à l'article 8 du projet de loi. D'autre part. Mais le problème qu'on a eu l'occasion d'évoquer à de nombreuses reprises en commission, c'est les flux de commandes. Et les livraisons des principaux matériels. Ne permettent pas pour l'instant de disposer d'une vision globale de l'exécution de la programmation militaire sur le plan pluri- annuel. Je rappelle que ce débat, nous l'avions eue sur la précédente LPM c'était la var la valorisation. Voilà. Valorisation actualisée. Des référentiels voilà et nous l'avions déjà introduit ça avait été voté et puis au moment de la CMP, nous avions été. Large d'esprit et nous l'avions supprimé. En revanche, nous tenons véritablement et ça a été exprimée. Par l'ensemble des groupes, et notamment des rapporteurs qui veulent effectuer un travail précis et conséquences sur l'état des commandes et des livraisons des principaux matériels plutôt que de disposer de d'informations éparses. Qui qu'on a parfois du mal à assembler on souhaiterait avoir la de PM qui nous permettrait d'avoir une vision d'ensemble peut-être sous forme d'un tableau mais un tableau vérifier et précis. Mais sur ce point je crois interpréter. L'ensemble la volonté de l'ensemble des groupes, pour avoir ce document de contrôle. Le Parlement est dans son rôle pour contrôler l'exécution de la programmation vous savez de quelle somme, il s'agit c'est parfois ce sont des milliards, il est quand même très important qu'on ait un oeil précis, année après année, sur ce sujet, donc évidemment nous émettons un avis défavorable sur la suppression de la communication de la de PM. Merci monsieur le rapporteur. le monsieur le Ministre, je je veux revenir sur ce qu'a dit Christian et je suis évidemment tout point d'accord lorsque. En 2018, on a demandé l'Avare. Cela fait tout hein. hein. Un cirque, on va dire ça comme ça et finalement le cabinet enfin décidée par par changer le nom. De manière à ce qu'on ne puisse pas en avoir la communication aujourd'hui, on estime que pour faire notre travail de parlementaire, on doit pouvoir bénéficier de l'apport que nous que nous donnerait la de dans un certain nombre de note. On nous dit que c'est trop compliqué qu'on n'y comprendra rien mais je crois que c'est à nous de juger finalement si c'est trop compliqué ou pas. Je pense qu'on a d'excellents élus et surtout d'excellents administrateurs qui sont tout à fait en capacité. d'étudier ce document donc moi je suis évidemment en en parfaite harmonie avec le président favorable à ce qu'on puisse avoir cette communication qui est importante pour nous qu'on ne réclame depuis 2017 et que par un changement miraculeux de non, on ne nous a toujours pas communiqué. Monsieur Perrin. Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement 243 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous avons 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Tout d'abord le 68 rectifié es mal. D'accord je vais pas je vous donner lecture

du projet de loi de finances, pardon des monnaies de financement des des matériels transmis donc voilà donc c'est c'est une marque de soutien bien sûr. Au peuple ukrainien qui se bat pour sa liberté donc là-dessus il y a pas de sujet nous conservons juste là aussi en terme de parlementaires, d'avoir la réalité du financement du matériel donc à passer a aussi quand on lit du matériel à pouvoir les retrouver aussi pour nos forces armées. Donc voilà c'est ce souci là que nous avons. merci madame la présidente. C'est effectivement un un amendement qui est issu notamment des qui avait été déjà déposé à l'Assemblée nationale depuis le début de la guerre en Ukraine, la France se fait un honneur de soutenir notre allié ukrainien face à l'agression de son voisin russe. Et si les prévisions sur l'issue du conflit sont incertaines. Mieux vaut prévoir le pire et l'inscription se confie dans le temps long. L'effort national de soutien à l'Ukraine et donc amené et là ça se prolonger dans le temps avec un financement adéquates. Aussi, il est essentiel que le gouvernement fasse la transparence sur le détail du soutien financier et militaire à accorder à l'Ukraine pour que le pas le Parlement puisse faire son travail de contrôle et juger de la suffisance. En ce qui nous concerne de ce soutien pour ne pas nuire à l'effectivité notre soutien en divulguant trop d'informations, cet amendement circonscrit la transmission de ces informations aux commissions compétentes des 2 assemblées via cette proposition d'amendement les groupes écologistes, nous souhaitons que le Parlement soit pleinement informé des détails de ce financement afin qu'il puisse exercer sa fonction d'examens et de supervision de manière rigoureuse. Depuis le début du conflit et malgré des consultations fréquentes via les débats 50 tirer hein. Le Parlement est trop tributaire des informations que le gouvernement veut bien du communiqué pour pouvoir se prononcer sur la poursuite de l'effort national associer le Parlement et obtenir son soutien informé c'est également consolider l'acceptation globale et sur le temps long de notre soutien au peuple ukrainien et nous le savons, l'issue de la guerre hésite pour beaucoup dans la capacité des pays occidentaux à maintenir leur soutien sur le temps long et au-delà des alternances démocratiques. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur. Avis de la commission sur ces deux amendements identiques. La présidente, c'est un avis favorable sur ces deux amendements identiques, en effet, il vise à renforcer. La transparence sur les modalités de notre aide l'Ukraine et les conséquences pour nos forces armées. Je rappelle que ces aides l'engagement du gouvernement ne doivent être imputée ni. Aux ressources budgétaires ni aux ressources extra-budgétaires, donc avis favorable. Si monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui. Le diable se nichant dans les détails. Moi je suis prêt à émettre un avis favorable à la mais avec un. Juste une demande c'est c'est sur un mot précis c'est de manière exhaustive. C'est le mot exhaustive pour tout un tas de raisons que vous comprendrez bien aisément. Exhaustif. Ça veut dire l'intégralité. Il est pas question évidemment de donner le signalement stratégique. À la Fédération de Russie enfin je pense que tout le monde le partage complètement et donc au fond il y a parfois, on peut dire qu'on donne un certain nombre d'éléments, on va pas forcément donner le nombre mais pour des raisons qu'on que vous comprenez aisément. Donc moi je ne vois plus sur le fond, il y a rien à cacher, en plus, vous le voyez bien en commission souvent je réponds à à à l'ensemble des des questions qui sont, qui sont posées en plus avec la la la la manière dont on a trié les dépenses il a Ukraine les dépenses ou les dons ne faisant pas l'objet d'un recomplètement exemple TRF1. Le milliard de dont on parlait tout à l'heure dans les 13 milliards je recommence pas. Mais qui touche au format des armées Crotale. AMX 10 RC 2ème catégorie 3ème catégorie le parc neuf hors LPM complètement les Césars bon en disant ça, des gens, on comprend un peu les logiques de moi je l'ai indiqué au président de groupe en tout cas ce que j'ai pu avoir et au président de commission. La prudence aussi de l'exécutif sur la soutenabilité de la LPM dans les années qui viennent. Elle passe aussi par cette évidence qu'il faut qu'on assume devant la nation. Ça a été dit par l'un et l'autre qui est que, évidemment, ce soutien. L'Ukraine va peser sur les finances publiques. Je crois que on l'assume, mais faut pas mentir évidemment à nos, à nos concitoyens, donc on a fait le choix que ça ne pèse pas sur le format des armées, donc ça ne pèse pas sur la LPM mais enfin il est évident quand on dit c'est hors LPM c'est quand même l'argent du contribuable qui va quand même de voir le nord et donc moi je suis évidemment favorable à ça donc moi proposition c'est une rectification des 2 amendements ou le mot exhaustif disparaît, ce qui me permet de garder une part de secret de discrétion sur certains aspects, je pense que vous pouvez complètement le comprendre en revanche que hélas dans la durée. Il y a une manière de notifier au président de commission. Ce qui l'aide à l'Ukraine. Je pense que ça va dans le bon sens et ça participera aussi à ce que toutes les sensibilités politiques prennent leurs responsabilités sur cette affaire, c'est assez gratuit. Ce que je dis ici. À l'Assemblée nationale avec une formation politique, ça l'était un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire, donc je pense que ça ça évidemment du sens on demande de rectification et si rectifier à avant. Merci monsieur le ministre. Alors si monsieur le rapporteur. On est d'accord et surtout si les auteurs sont d'accord pour rectifier leurs. Leurs amendements en supprimant de du 1er membre de phrase hein de l'alinéa. Qui diraient les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informés, on supprime de manière exhaustive et on poursuit effectivement la rédaction de La Linea si nos 2. Auteurs sont d'accord et si monsieur le rapporteur. Vieux bien nous donner son avis. Le rapporteur et d'accord sur cette rectification qui a été fait dément tout à fait utile. Très bien. Alors je vous propose de mettre aux voix les 2 amendements rectifiés qui deviendraient les 68 rectifié bis et 139 rectifier quater donc modifier et supprimant de manière exhaustive, je les mets aux voix avec un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour.

Il est adopté. Article additionnel après le 9 bis. 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 156 rectifié c'est monsieur Laurent qui le présente. Monsieur le président. Merci madame la présidente. Il s'agit d'un amendement sur le contrôle des des ventes d'armes, nous avons des des. L'an l'an dernier une proposition de loi assez complète sur le sujet. Je crois que c'est un sujet qui est maintenant récurrent et qui appellent des progrès dans les garanties démocratiques et de la transparence significatif. La France et 3ème. On parle même maintenant de. 2ème rang exportatrice mondiale d'armement. Mais nous sommes très en retard du point de vue des garanties démocratiques et de la transparence. Contrairement à de nombreux parlements. Européen mais pas seulement. Dans lequel il existe des commissions parlementaires dédiée chargée de suivre de près les contrats d'armement. Non, nous proposons un dispositif qui est de créer une délégation parlementaire. Interparlementaire chargée de contrôler les autorisations et les licences qui disposeraient si nécessaire. D'un droit de véto dont les travaux seraient couverts par le secret de la défense nationale. Les dispositions que nous proposons sont plus ambitieuse. la l'amendement que que présentera. Tout à l'heure le président Cambon. Sur le même sujet visant à charger la délégation parlementaire au renseignement de cette. Mission. Je pense qu'il faut que nous progressions significativement sur ces questions, d'abord pour des raisons démocratiques pour des raisons de de de contrôle de la destination de ces armes, mais aussi pour une autre raison c'est que. Nous installons un modèle de base industrielle technologique de défense qui est. Organisé autour de l'ambition d'exportation et et donc tout ça appelle des contrôles beaucoup plus sérieux qu'ils ne le sont aujourd'hui par le Parlement. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sérieux par les commissions. Dédiées qui s'en occupe mais en tout cas le Parlement lui n'a pas les moyens de ce contrôle sérieux et donc voilà pourquoi nous faisons cette proposition.

qui à peu près identique hein et qui s'appuie sur les propositions formulées par ce maire Tabarot dans leur rapport d'information sur le contrôle des exportations d'armements, ainsi que sur les travaux d'Amnesty International et du Parlement européen. De nombreuses propositions de loi à ce sujet ont par ailleurs et tu as déjà déposé à l'Assemblée nationale et au Sénat par différents groupes politiques, ce qui témoigne justement d'un constat transpartisan et évidemment de la nécessité de renforcer le contrôle du Parlement en matière d'exportations On pas reprendre tout ce qui vient d'être dit précédemment, pense que l'instauration d'une délégation parlementaire permettrait au Parlement d'effectuer un contrôle a posteriori efficace de la politique d'exportation d'armements et de biens à double usage de la France ainsi que de s'assurer. Que les décisions respectant les engagements internationaux de de la France en matière de droit humanitaire, tout en respectant évidemment le secret défense. Merci.

qu'il est normal que le Parlement dans ce rôle d'évaluation de des politiques publiques et cetera puissent avoir accès. Donc c'est bien cette logique d'évaluation a posteriori. C'est dans un cadre bien sûr de secret défense. Donc c'est ça notre, notre proposition en sachant que on va regarder également l'avis qui sera donné sur l'amendement 293, conformément à l'engagement qu'ils ont pris puisque je crois que et je l'ai dit d'ailleurs au ministre et et au président. À force de ne pas avancer. On passera un jour de rien, ce que nous sommes aujourd'hui à un contrôle total même avant même de vendre et donc la proposition qui nous est qui qu'on vous fait nous c'est d'avancer la logique des petits pas, il vaut mieux progresser avec cette logique d'évaluation. Via le secret défense plutôt encore une fois de faire laisser monter les enchères. Jusqu'au jour où ne pourront plus faire autrement que d'avoir une une un contrôle a priori. Merci cher collègue. Le 200 a rectifié Monsieur Gontard. madame, madame la présidente. Cet amendement est un repli par rapport au précédent, il était également inspiré par Amnesty International et les travaux du Parlement européen. Et plutôt que de créer une nouvelle délégation parlementaire, il vise à étendre le Champ de compétence de la délégation parlementaire ou saignements pour pouvoir y ajouter des prérogatives relatives à l'exportation d'armements et des biens à double usage, ce n'est pas forcément l'option privilégiée par le rapport de nos collègues. Jacques Maire et et Michèle Tabarot, qui lui préfèrent des solutions plus en 2 BBC eux mais nous semble être une possibilité de trouver un compromis, la délégation parlementaire ce étant soumise au secret défense. Cela permettait notamment de conjuguer un minimum de contrôle parlementaire avec les exigences, lourdes, parfois même trop lourde du secret défense. L'extension des prérogatives de la DPR est également le choix qu'a fait notre rapporteur, et je salue au passage ce soit fort de la majorité sénatoriale qui permettrait enfin la France de se conformer au code de bonnes pratiques de l'Union européenne dont l'importance a été rappelé par des résolutions du Parlement européen de 2008 et de 2021. C'est vrai que la, la mouture du de l'amendement qui suit justement de la de la commission. Nous sommes d'ailleurs plus intéressantes que cet amendement puisqu'elle crée une commission au sein d'allégations parlementaire aurait seulement avec quatre parlementaire dédiée à ce sujet. Donc ça me paraît plus. donc soit on rend notre amendement identique à celui d'après, ou en tout cas on votera le 293. Merci. Merci Monsieur Gontard enfin le 293 monsieur le rapporteur. Au nom de la commission des Affaires étrangères. Alain présidente. Nous sommes là sur un, un sujet important qui revient régulièrement dans les questionnements que se pose le parlement au sujet du contrôle des ventes d'armes. On sait que c'est un sujet qui est dans d'autres parlements qui fait l'objet de. 2 contrôles beaucoup plus. Importants que ce que nous connaissons. Quelle est la situation à l'heure actuelle. Les ventes d'armes font l'objet d'un examen par une commission présidée par le Premier Ministre là siège et qui examine les licences d'exportation et qui selon des critères qui sont tout à fait. Bien Bien identifié. Émet un avis favorable ou défavorable. Sauf que. L'ensemble de ce travail ne donne lieu qu'à un assez modeste, rapport, il a été, je veux dire sous sous. Grâce à vous, du reste il a été un peu épaissie ces derniers temps mais il ne permet en aucun cas un véritable échange politique comme on doit l'avoir, dans un régime parlementaire ou les ventes d'armes. D'un pays comme le nôtre qui est quand même cela a été cité. Un, un des pays pointe dans ce domaine et qui. Est sous-tendue par 200.000 salariés qui travaillent par nos, pour nos industries d'armement, donc ce n'est pas un problème tout à fait négligeable mais donc ce ce contrôle et cet échange politique. Ne peuvent pas avoir lieu. Il est assez normal que des que différents groupes se soient manifestés au sein de la commission pour faire des propositions qui ont été examinés et moi-même je me suis engagé au cours de la commission a déposé un amendement qui n'est pas totalement inconnu puisque en fait il faisait l'objet d'une proposition du PPL qui à l'époque je ne je n'avais pas je n'avais pas défendu, même si j'avais reçu les encouragements du Ministre de la défense de l'époque. En l'occurrence de quoi s'agit-il. Il s'agit d'utiliser un organisme que nous que vous connaissez bien, au moins par le nom, la délégation parlementaire au renseignement qui est un organisme inter-parlementaire, c'est-à-dire qui rassemble 4 députés et 4 sénateurs. Qui travaille bien évidemment à contrôler. Les activités de renseignement y compris du reste avec une sous-commission chargée du contrôle des fonds secrets. Cette commune ce cette délégation fonctionne depuis 10 ans à la plus grande satisfaction des gouvernements successifs puisque. Les règles qui s'imposent. Aux membres de cette commission j'en suis il y en a d'autres ici notamment le président Buffet qui a présidé aussi cette DPR puisqu'il y a une alternance, assemblée nationale, Sénat pour la présider cette commission. Travail depuis 10 ans et a toujours strictement respecté les conditions extrêmement sévères qui nous sont imposées de secret absolu. Il y a pas de téléphone, on est dans une salle blanche et on on remet hein on on auditionne bien évidemment les personnalités que l'on souhaite entendre sur des problèmes de de de renseignements. Imaginez ce qui a pu être le cas au moment du terrorisme. Bien sûr, les activités de des actions de terrorisme et puis la DPR remet un rapport. Circonstancié au président de la République, c'est un rapport dont le président de la République après fais j'allais dire ce qu'il ce ce qui lui en veut. C'est-à-dire qu'il peut enlever retirer faire retirer des éléments. Qui ne doivent pas de son point de vue être communiquée au public et donc cet organisme fonctionne, il existe, il est très apprécié et il n'a jamais porté atteinte aux règles de fonctionnement et de secret que j'évoquais il y a un instant et donc plutôt que de créer des délais une délégation nouvelle avec tout ce que la tout J'ai pensé pour ma part qu'il était plutôt utile d'utiliser cet organisme. La délégation parlementaire au renseignement et y créer une sorte de commission exactement à l'image de la commission de vérification des fonds spéciaux, une commission qui vérifierait les a posteriori bien évidemment les exportations d'armes concrètement comment les choses peuvent se passer. Le rapporteur de la sienne, je peux venir une ou deux fois par an dans une séance spécifique devant cette sous-commission rapporté à la fois les les les résultats en quelque sorte les autorisations de licence et les refus de licence de telle sorte que le gouvernement puisse si il est attaqué et il le sera un jour qu'un jour, un jour il y aura fatalement un accident qui sera déplorable et il pourra dire j'ai rendu compte de mon activité au Parlement et le Parlement pourra dire qu'il a effectivement entendu. Le gouvernement et qu'il a fait rapport au président de la République lequel et de par ses compétences. Tout à fait. En mesure de prendre des décisions qui s'imposent. Voilà pourquoi nous pensons que cet cet amendement peut se substituer, avec le soutien de de mes collègues qui ont déposé les autres amendements qui sont tout à fait respectable et qui vont tout à fait dans le même sens mais je supplie le gouvernement de nous entende sur ce sujet de très nombreuses ONG de très nombreux journalistes suivent les activités de vente d'armes de la France, vous le savez. un jour ou l'autre. Lorsqu'il y aura un problème ou même s'il n'y a pas de problème. Un jour ou l'autre il faudra bien trancher ce sujet, il y avait eu une ouverture qui avait été fait par l'ancien 1er minis Jean Castex je lui rends hommage il avait autorisé par voie de décret. L'autorisation à 3 ministres, celui des armées celui des affaires étrangères et celui de l'Économie et des Finances, de venir nous rencontrer ensemble devant le bureau ou devant une formation de de chacune de nos assemblées mais jusqu'à présent, les 3 ministres n'ont pas pu trouver le temps mais on sait que leur emploi du temps est très chargé pour se rendre à ses convocations que du reste. Nous n'avons pas. Renouvelé puisqu'on n'a jamais réussi. À avoir un feu Vert pour réunir cette ce qui ne correspond pas du tout au sujet en quelle que sorte que nous venons d'évoquer. C'est pour ça que l'utilisation de la DPR nous paraît être. Une bonne occasion de régler une bonne fois ce problème et de faire un pas qui à mon sens s'arrêtera là. Mais il sera quand même très utile pour le contrôle parlementaire. Si monsieur le rapporteur. Donc on en déduit, bien que vous demander le retrait des 4 amendements au bénéfice du 293. de ces groupes, il y a déjà des membres qui ont siégé ou qui siègent au sein de la ADP. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Défavorable. Je vous remercie. À l'ensemble des amendes mais on est bien d'accord. Alors monsieur tu d'abord. Nous regrettons que le gouvernement dit juste. Un mot et pas plus je pense encore une fois. Comment. Si si ça sert il y a des sujets là il y a fait qui servent je je le redis, mais comme l'a dit le président quand bon c'est un sujet qui est et. Qui est éminemment important et je crois encore une fois que l'évaluation est nécessaire sinon il y a un moment donné on passera à une autre logique, enfin quand on dit nous,

et par la la délégation et donc c'est pour ça que nous retirons notre notre amendement au bénéfice effectivement de l'amendement 293, déposé par le rapporteur. Merci. Bon, la réponse lapidaire de Monsieur le Ministre, qui depuis le début de notre débat était quand même assez disponible pour répondre aux questions et n'est n'est pas très Sur un sujet qui manifestement. Qui a gagné beaucoup en sensibilité toutes ces dernières années et si il y a des amendements venus de hiver à une proposition du président de la commission. Je pense que ça mérite un peu plus d'égards sur un sujet qui, sinon on va continuer à monter dans cette situation nous comme nous ne sommes pas des partisans du tout ou rien, même si nous avons déposé des propositions parlementaires nous allons retirer notre amendement au profit de l'amendement du président quand bon même si nous jugeons la proposition encore timide mais au moins expérimentons le dispositif. Que préconise le président de la commission et et nous aurons au moins une première. Possibilité d'agir et puis ensuite, nous verrons si ça suffit ou si ça suffit pas mais avançons. Si cher collègue, et donc au retrait de l'amendement 156 rectifié au bénéfice du 293 le Monsieur Gontard pour. Explications de vote. Et merci merci madame la présidente. de la manière, c'est vrai que je, je regrette effectivement à la fois le le manque d'explications du du du mini-sur cette, cette décision est sur quand même le le travail qui a été qui a été fait par la commission pour arriver à trouver ce ce compromis et qui me paraît plutôt. Plutôt assez juste donc je retirerais 199 après je crois le, le 200 très très proche du 293 donc si je peux le rectifier pour rendent identique aux 293 voilà. Il est rectifier. Donc c'est le 200 hein qui devient un amendement rectifier identique au 293. De la commission. Donc ça devient un rectifier bis 200 hein et donc je vais mettre aux voix avec un avis favorable du gouvernement. Les 2 amendements identiques.

Les comptes. Qui s'abstient. Ces deux amendements sont donc adopté. Oui. Ensuite, je mets aux voix l'article 10. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il était adopté. On il y a un article 11 qui s'est caché derrière. Donc, je veux voir l'article 11. Même avis même vote même vote après l'article 11, un amendement 32 rectifié. Monsieur Guillaume. Qui n'ont pas pu bénéficier d'une allocation de reconnaissance du fait de la distinction après la guerre d'Algérie entre les supplétifs de statut civil de droit local et ce de droit commun. Dans ce cadre, les premiers ont bénéficié de l'attribution d'une allocation spécifique de reconnaissance. Par sa décision du 4 février 2011. Le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relatives au règlement de l'indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun. Également éligible à l'attribution de l'allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011. J'espère qu'on m'avait suivi en réponse à cette ouvert la loi du 18 décembre 2013 relatives à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a finalement réservé cette allocation aux seul supplétifs de statut civil de droit local cependant dans cet intervalle tous les supplétifs ayant formulé une demande de renouvellement de demande, entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation. Aujourd'hui ils ne sont plus qu'une vingtaine à espérer. Cette mesure de réparation d'un montant de 4150 euros. La commission a introduit cette question au sein du rapport annexé de l'article de toutefois mon groupe a souhaité qu'elle soit évoqué en séance publique. Bien entendu il s'agit de l'amendement d'appel puisque compte tenu des règles de recevabilité financière. Il est ici prévue à défaut de pouvoir créer la location d'exonérer d'impôt sur le revenu. Les membres de ces formations supplétives. Sans méconnaître le fait que la situation fiscale des personnes visées de permettra sans doute pas de leur donner satisfaction. Je souhaiterais aussi, Monsieur le Ministre rappeler que le Sénat s'était déjà prononcé 2 fois favorablement sur ce sujet lors de l'examen des lois de finances de 2019 Merci cher collègue. des supplétifs de droit commun à qui nous devons encore longtemps après les événements. Une véritable reconnaissance et cet amendement vise à donc à exode les inexorable des impôts sur le revenu. Alors malheureusement, il est assez difficile d'évaluer ce que cette exonération représenterait pour les personnes en particulier notamment certains de ces supplétifs ne sont vraisemblablement déjà pas soumis à l'impôt sur le revenu et en commission, nous avons préféré adopter l'amendement du président Laurent qui a été présenté au nom du groupe communiste. Et qui sera dans le rapport annexé et qui prévoit une indemnisation forfaitaire de 4195 euros par supplétifs et ce dispositif nous paraît nettement préférable donc soit retrait soit un avis défavorable sur cet amendement. Merci monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. À du gouvernement. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Carrère. Le gouvernement est attaché à ce que les mesures fiscales soient examinées dans le cadre des projets de loi de finances. par conséquent je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement mais sur le fond pour répondre. À vos à vos interrogations. Sinon il y a pas lieu de prévoir un régime fiscal particulièrement dérogatoire pour les harkis blanc cela poserait une difficulté au regard du principe d'égalité. Je rappelle que la situation des harkis blanc doit être assimilée à celle des autres rapatrie européen. Et ne peut, à ce titre, considérer qu'ils ont subi un traitement défavorable justifiant l'octroi d'une allocation ou d'un Avantage fiscal à leur arrivée en France, ils ont en outre perçu les mêmes aides, à savoir des prestations temporaire de subsistance des subventions d'installation des prêts à taux réduit. Des aides de reclassements professionnels des secours, et c'est Lionel donc je je je mettrai un avis défavorable.

Merci cher collègue. Il est donc retiré, c'est le 32 rectifié. Après l'article 11, nous avons un amendement 38 rectifié monsieur Cabanel le défend. Merci madame. La présidente Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Mes chers collègues. Tous les jeunes appelés à leur journée de défense et citoyenneté se voit dispensé plusieurs heures d'enseignement au fil du temps le contenu de cet enseignement désormais inférieur à 3h s'éloigne de plus en plus du coeur de cible de cette journée. En effet, outre les enseignements initiaux concernant les âges à la défense nationale au sens large des modules ont été intégrés au gré des évolutions de la société par exemple une information consacrée à l'égalité entre les femmes, les hommes à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple a été intégré au programme à partir de l'année 2020. Une autre information concernant la prévention des conduites à risques pour la santé avait été inséré à compter de juillet 2016. Ça bien entendu vouloir minimiser l'importance de ces, de ces sujets la JDC au regard de sa durée limitée, ne peut pas tout transmettre par conséquent cet amendement vise à se recentrer à recentrer la journée de défense et citoyenneté sur les priorités suivantes l'information sur les enjeux de la défense et de la sécurité et sur les métiers accessibles aux jeunes dans ce domaine. Le repérage et l'orientation des jeunes en difficulté, conformément, une volonté exprimée par le législateur en 1997 lors de la suspension de la conscription de favoriser l'aide à l'insertion et enfin la présentation des différentes formes d'engagement que sont notamment le service civique. Le volontariat, la réserve ou encore la sécurité civile. Cette nouvelle rédaction maintiennent naturellement les tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française qui préfigurait déjà au programme de la journée d'appel de préparation à la défense. Merci cher collègue monsieur le rapporteur. avec le rapport d'information qui s'intitulait jeunesse et citoyenneté une culture à réinventer qui avait été adoptée par le Sénat en juin 2022. Je rappelle que le programme de cette Journée défense et citoyenneté a été modifiée 12 fois par le législateur. Entre 2000 et 2021 et que le temps consacré aux questions de défense, comme l'a dit notre collègue était inférieur à 3h. Donc je pense que les problèmes de défense doivent être mieux présentés afin de sensibiliser nos jeunes et donc c'est un avis tout à fait favorable.

En fait il y a une étude qui est en cours pour recentrer la JDC sur l'enseignement de défense car il y a un enjeu fort de recrutement pour les armées. La JDC constitue une formidable occasion de de faire connaître la défense et ses missions comme elle. Constitue aussi l'occasion unique de toucher l'ensemble d'une classe d'âge. Des travaux sont en cours pour trouver une autre voie pour atteindre le résultat que vous recherchez à travers la LPM, nous réfléchissons à consulter le Conseil constitutionnel pour qu'il constate le caractère réglementaire des dispositions actuellement en vigueur, nous permettant ainsi de les modifier par voie de décret en Conseil d'État. Voilà donc j'espère vous avoir convaincu Monsieur le Sénateur Cabanel. Merci madame la ministre. Alors monsieur Cabanel, vous voulez prendre la parole pour explication. J'ai juste pour. Remercier Madame la Ministre de ces explications. Je ne doute absolument pas de sa parole bien entendu mais bon pour avoir assisté comme comme pas mal d'entre nous a a séjourné 2 défaillent seule citoyenneté je je je pense quand même qu'il est nécessaire même si vous avez l'intention de le faire, je vais quand même maintenir on amène demain. Si cher collègue. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 38 rectifié qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Et nous avons maintenant un amendement 245 monsieur le Madame la Ministre du gouvernement décidément. Peut être madame la présidente, vous dire que je vais défendre les amendements jusqu'au 249. c'est un amendement du gouvernement qui vise à lever les seuls pupille de la nation. La forclusion opposable depuis 2018 à toute demande de pension en raison d'actes de violence subie lors du conflit algérien. Il s'agit d'accorder une reconnaissance pleine et entière à ces quelques dizaines d'orphelins personnellement blessés au cours de la guerre d'Algérie en leur rouvrant la possibilité de prétendre à une pension civile de guerre. Je vous précise que cette demande sera toutefois limitée dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la LPM. Merci madame la ministre monsieur Cambon avis de la commission sur le 245. Alors ce sera un avis favorable et car cette mesure de reconnaissance est la bienvenue pour des personnes qui ont été victimes du conflit algérien et qui était étrangement exclus depuis 2018 du dispositif, alors que plusieurs dizaines d'entre eux blessé pendant la guerre d'Algérie n'avait pas pu en bénéficier. Avis favorable. Merci monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement 245 qui a reçu un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté, Il y a 2 amendements et un sous-amendement qui font l'objet d'une discussion commune et nous commençons donc par le 55. Merci madame la présidente Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement procède à la modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre le sous l'acronyme connu Afin de compléter notamment l'émission de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, plus connu sous l'acronyme ONAC VG. Stratégiquement, vous comme vous le savez, mes chers collègues, l'Office sera confrontée dans le rôle de relais territorial de l'action mémorial du ministère qui était animé par la direction de la mémoire de la culture et des archives du ministère des Armées. Donc cet amendement consiste de manière relativement succincte à insérer un article additionnel ainsi rédigé l'Office concours à la mise en oeuvre de la politique de la mémoire combattante défini par le ministre chargé de la défense pour inclure le le sous-amendement du gouvernement qui suit. De l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Merci. Monsieur le nez le défend. Oui. Mais, présidente. Madame la Ministre, Monsieur le ministe cet amendement procède à la modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour compléter l'émission de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. La mission de l'Office sont pour l'essentiel, centré sur les droits des ressortissants. Or l'ONAC. Largement développé depuis plusieurs années des actions mémorielles de grande qualité à destination notamment de la jeunesse. Au-delà de sa mission. L'Office s'est en effet particulièrement investie dans le Patrimoine mémoriel de Pierre nécropole nationale et au lieu de la mémoire nationale, justifiant ainsi son action dans le Champ de la mémoire combattante et stratégiquement le fils sera conforté dans son rôle de Rola territoriale de l'action mémorial du ministère qui est animé par la direction de la mémoire de la culture et les archives du ministère des Armées. Y'chers collègues. Nous passons à la présentation du sous-amendement 289 présenté par le gouvernement. Madame la ministre. Alors il s'agit d'un amendement rédactionnel puisque l'ONAC qui était et étant placée sous la tutelle du ministre de la Défense au terme de l'article L 611 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. Il convient de modifier l'alinéa IV qui fait référence au ministre chargé des Anciens combattants. Par de la Défense. Voilà dans la mission mémoriel confiée à l'Office. Donc je je veux je vous donnerai même un avis favorable pour les 2 amendements précédents à condition que le rédactionnel soit votée. Merci. Merci. Si madame la ministre et donc monsieur le rapporteur. Votre avis sur cet ensemble d'amendements et le sous-amendement. Je suis à ma présidence, j'ai commencé par le sous-amendement de 189 bien évidemment. Un avis favorable a qui est en effet bien sous la tutelle du ministre de la Défense et un avis favorable au à l'amendement 55 et aux 113 rectifié bis car effectivement c'est une très bonne initiative d'ajouter la mise en oeuvre de la politique. De mémoire de la mémoire combattante à le ONAC tout ça va exactement dans le bon sens. Avis favorable. Merci monsieur le rapporteur. Madame la Ministre ou souhaité reprendre la parole. Oui parce que je voudrais profiter de ces amendements pour. Pour saluer saluer l'action décisive des femmes et des hommes de l'ONAC départemental qui font un travail formidable sur nos territoires et donc ça me donne l'occasion de les remercier. Dire aussi que. L'ONAC Fillon-travail formidables sur les hauts lieux de mémoire sur les nécropoles sur l'arme leur entretien et et sur la conservation évidemment du souvenir des combattants français je me suis engagé aussi avec les actions les associations dans le sien combattant pour la jeunesse parce qu'il est important de montrer à notre jeunesse et au lieu de mémoire. Donc je me suis engagé parce que la déco, la décentralisation de certaines commémorations nationales. Que je souhaite faire chaque année qui tourneront selon les années. Comme je l'ai fait à notre dame de Lorette, le 19 mars où il y a eu 400 personnes avec 200 jeunes je l'ai fait aussi au Struthof. Il y a eu 300 personnes avec 180 jeunes et je l'ai fait à nouveau. Au mémorial d'Indochine à Fréjus nous avons aussi vu 200 jeunes sur c'est au lieu de mémoire. Donc voilà c'était pour vous dire que nous avons travaillé avec les associations d'anciens combattants pour faire tourner un petit peu et aller vers vos territoire puisque je pense que c'est important de venir aussi montrer ce que vous faites tous les jours et ce que fait l'ONAC sur les territoires. Merci. Merci madame la ministre et j'de demandes d'explications de vote monsieur Folliot. Vous avez la parole, cher collègue. Oui merci madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Bien entendu, je soutiens ces amendements puisque je ne suis co-signataire et ainsi que le sous-amendement. Du gouvernement mais je voudrais simplement dire que au-delà de l'ONAC. Je voudrais attirer l'attention de la. Du du Sénat sur le rôle du Souvenir français qui est une association qui a des missions qui sont aussi dans ce cadre-là, qui est tout à fait exemplaire. Avec des bénévoles avec un maillage territorial assez somme toute. Important au niveau national et je crois qu'il me paraît important de le dire ici et de veiller à ce qu'il y ait une bonne et saine complémentarité entre. Ses missions de l'ONAC élargie et celle du Souvenir français parce que je crois que il y a un enjeu qui est un enjeu important pour finalement qu'on vous l'avez dit Madame la Ministre perpétrés cette mémoire combattante, qui est un enjeu essentiel mais aussi faire tout ce travail de l'ombre et qui consiste souvent à aller sur les carré militaire à restaurer des tombes à faire tout ce cet important. Travail visant à essayer de sauvegarder des pans entiers de notre mémoire combattante qui. Sont en train. Finalement, au fil du temps de nous quitter et je crois que c'est

Oui merci. Merci. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre je tenais aussi à. Témoigner et soutenir ces amendements bien entendu que je suis soutiendrez

le rapport d'information remonte à. Octobre dernier sur l'ONAC en tant qu'opérateur de l'État et donc. Vous êtes notre interlock bon interlocuteur concernant, et je parle au nom des collègues de la commission des finances sur la mission. On tient combattant lien avec la nation et et mémoire avec 2 opérateurs de l'État l'Institution nationale des invalides et l'ONAC. ONAC VG, on dit toujours mais je dirais on est.

au monde combattant aux associations patriotiques et de mémoire et l'ONAC est réellement à la disposition du monde combattant et puis le lien avec la jeunesse. Vous l'avez rappelé, madame la ministre, je crois que c'est réellement fondamental et le maillage du territoire. Tous les départements. Métropole, Outre-mer et Afrique du Nord. Je crois que justement l'ONAC. C'est aussi hein. C'est un combat permanent de de maintenir 3 4 personnes ou 5. Par département pour être à la disposition du monde combattant. Donc je suis soutiendrai bien entendu ces amendements, merci. monsieur Laménie. Alors je vais mettre aux voix le sous-amendement du gouvernement numéro 289 qui a donc un avis favorable de la commission. Donc il est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il est adopté et je mets donc aux voix maintenant les 2 amendements identiques ainsi sous-amendé le 55. Et le 113 avec donc un avis favorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils sont adoptés. Après l'article. Le 11, nous avons le 244 qui est présenté donc par le gouvernement Madame la Ministre. Merci madame la présidente, la préservation et la mise en valeur du Patrimoine militaire. Contribuer au renforcement du lien entre la nation et son armée. Il est souhaitable que le droit positif en matière de cession et de mise à disposition de bien à titre gratuit évolue afin de rendre pleinement effectif ces mécanismes et développer des partenariats avec les collectivités territoriales et les associations en ce domaine. Ainsi le présente un amendement vise à permettre la mise à disposition à titre gratuit des biens meubles dans le ministère de la Défense n'a plus emploi aux seules associations et organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du Patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la nation et son armée supprimer le plafond limitant le mécanisme de cession à titre gratuit de c'est bien dans les seuls cas où les sessions ont pour destinataire de telles associations. Je précise que les les cessions de biens ou matériel ne donne pas droit à une mise en vente évidemment de ses biens. Merci madame la ministre, monsieur le rapporteur. La présidente de c'est un avis favorable de la commission, je pense que ceci va dans le bon sens, je précise bien qu'il s'agit des biens meubles comme par exemple ceux-ci va permettre la session plus fluide d'aéronefs de collection à des associations qui mettront en valeur le Patrimoine militaire. Avis favorable. Je mets donc aux voix l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission. Qui est pour. Qui compte. Qui s'abstient il est adopté le audit. Alors. Ces deux amendements qui sont en discussion commune le 202 rectifié Monsieur Gontard. Arbitrairement condamné à mort et fusillé pour l'exemple, pendant la Première Guerre mondiale pour des eaux Byzance militaire il reprend notamment la proposition de loi de notre collègue Bastien Lachaud adopté à l'Assemblée nationale est rejeté par le Sénat en janvier après un riche débat depuis février, la majorité sénatoriale qui s'inquiétaient d'une réécriture de l'histoire nous a proposé à l'adoption du Sénat de propositions de résolution pour reconnaître le génocide assyro-chaldéens de 1917 et 1921 et de reconnaître la grande famine de l'eau de mort comme une entreprise génocidaire face à cette nouvelle disposition de la majorité de réinterroger la mémoire des nations. Je me permets donc de poser à nouveau le cas des fusillés pour l'exemple de la Grande Guerre. Le présent amendement vise à réhabiliter ses 639 soldats et conclure ce travail mémoriel engagé au Parlement dès 19.116. À la fois par Lionel Jospin et Nicolas Sarkozy. Sarkozy plus récemment. Il s'agit ici de rassembler la nation en réparant tant bien que mal les injustices commises à la con de ces fusillés, dont les souvenirs restent très vif, notamment au sein de leur famille. Merci. Merci cher collègue guère le 152 madame Gréaume. Merci madame la présidente. La question des fusillés pour l'exemple est une question qui tient à coeur mon groupe et je tiens d'ailleurs à rendre hommage à l'ancien sénateur Guy Fischer qui avait porté avec brio cette question dans l'hémicycle. Effectivement, le groupe communiste et citoyen à l'époque avait déposé en 2013 une proposition de loi visant à répondre à la demande juridique et mémorielles au sujet de la réhabilitation. Notre amendement vise donc à réhabiliter l'ensemble des soldats, fusillés pour l'exemple, durant la première guerre mondiale. En effet, nous considérons qu'il n'est pas possible de faire le tri. Plus de 100 ans après, entre les soldats, fusillés à tort, victime de condamnations arbitraires ou abusive et ce dont l'exécution était justifiée l'adoption de cet amendement sera un acte toute fraternité pour la mémoire de ces hommes qui furent jetés dans l'arène meurtrière des tranchées et qui furent vaincus par l'épuisement. Alors, mes chers collègues sachant aujourd'hui qu'il n'y a plus de témoins. Et que notamment beaucoup de preuves sont en partie détruites. Je vous demande d'y réfléchir. De nombreuses associations le réclament ainsi que la Ligue le de la Ligue des droits de l'homme. Donc aujourd'hui il est temps de le rendre ce qu'il faut c'est de réhabiliter les fusillés pour l'exemple. Merci Madame la présidente. Il s'agit d'un sujet d'une très grande gravité mais aussi d'une grande complexité qui vous le, vous vous en souvenez, a fait l'objet d'une discussion ici, en première lecture en février dernier et qui a été rejeté. Par le Sénat et donc en cohérence avec ce que le Sénat a décidé il y a quelques mois je propose. Un avis défavorable pour ces deux amendements en discussion commune. Merci madame la ministre avait du gouvernement. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Gontard, madame. Gréaume. Je je vais redire ce que j'ai dit le 2 février. Ici, ici même au moment du passage de la LPM fusillés D'abord votre proposition heurte le monde combattant, notamment sur l'inscription des noms. Sur les monuments aux morts depuis la première guerre mondiale, les assemblées par parlementaires ont déjà battu débattu. De loi d'amnistie et de révision leurs conclusions a toujours été la même à une condamnation individuelle ne peut répondre. Aucune réhabilitation individuelles. En effet, la réhabilitation générale poserait problème si certains fusillés pour l'exemple, ont été condamnés à l'issue d'une justice militaire expéditive. D'autres l'ont été à raison de crimes qui ne sont pas pardonnable. C'est la raison pour laquelle la réhabilitation doit demeurer du ressort de la justice toute réhabilitation générale empiéterait sur le principe de séparation des pouvoirs. Votre amendement semble méconnaître le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Je vous propose donc de retirer cet amendement dans le sujet n'a pas de lien avec la LPM, merci. Merci madame la ministre. Il n'y a pas d'explication de vote. Je vais donc mettre aux voix, pardon monsieur Laurent, excusez-moi. Ce sera très court mais je trouve les deux réponses qui sont faites et singulièrement celle de la ministre désolante d'inhumanité sur ce sujet.

doit avoir lieu à l'aura lieu donc autant qu'elle se fasse le plus rapidement possible. Madame la Ministre, vous souhaitez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, Laurent, je ne peux pas vous laisser dire ça. J'ai une attention particulière depuis le 4 juillet. Depuis que j'ai été nommé. Nous avons eu ici les discussions. J'ai expliqué, je ne sais pas combien de fois que on ne peut pas faire une réhabilitation de de. Il faut qu'elle soit individuelle, il y a dans les archives, la possibilité, et ça a été fait d'ailleurs ça a été fait il y a des fusillés, qui ont retrouvé je vais dire l'honneur. Et donc ce que je vous invite à faire et je l'avais déjà dit c'est de regarder dans les archives. Je suis désolé, il y a des familles qui l'ont fait, donc vous aurez bio remettre je vous ai donné l'explication, ce n'est pas possible. Ici nous sommes dans un dans une assemblée et ne ce n'est pas la justice. Donc vous comprendrez que ce n'est pas possible. Merci je vais mettre aux voix l'amendement 202 rectifié qui a reçu 2 avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. S'abstient. Il n'est pas adopté le 152 rectifié même avis même vote. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix. L'article 11 bis. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Et le 11 bis, un amendement 51. Ratifier. Qui le défend le 51 rectifié. Monsieur Burgot. Ah il est défendu. Le. Il est défendu avis de la commission. Monsieur le rapporteur. c'est un avis favorable. Madame la présidence pour un amendement qui propose de rendre enfin possible l'inscription du nom des militaires morts pour la France sur le monument aux morts de la commune où ils sont inhumés auparavant ce n'était pas possible et donc c'est un avis favorable cet ajout permettra que leurs noms figurent sur le monument de la commune où ce soldat repose. Merci monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur du roi, alors évidemment c'est un avis très favorable. Très favorable parce qu'il permet aussi de réaffirmer le lien mémoriel entre les territoires qui sont tombés. Pour la nation, mais surtout aussi de répondre à un souhait des familles. Alors je vais répéter parce que peut-être vous avez pas entendu le souhait des familles et je crois que c'est c'est pas grave. Monsieur Retailleau. Mais voilà et je pense que c'est ce que on doit aussi aux familles de de ces morts pour la France et donc c'est des. Je me répète, mais c'est un avis très favorable. Merci. Merci, madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 51 rectifié qui a reçu 2 avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il était adopté. Amendement 189. Madame Garriaud-Maylam Oui merci beaucoup madame la présidente. Il s'agit de bien réaffirmer le caractère impératif des journées de défense et de citoyenneté pour les jeunes. Français de l'étranger. J'ai déjà au lit, eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet dans la discussion générale. Il est impératif que ces jeunes qu'ils soient mono-nationaux français peut être plus encore s'ils sont binationaux puissent avoir accès à une connaissance de ce qu'est notre outil de défense de nos enjeux géostratégiques donc en introduisant la notion, sauf circonstances exceptionnelles cela permettent de montrer combien il est important d'organiser Cegid. Pour les Français de l'étranger. Pour mémoire, il avait été décidé par le Quai d'Orsay de les supprimer tout bonnement pour soi-disant des raisons budgétaires. ceux-là est évidemment inadmissible dans la mesure où en plus cela ne coûte quasiment rien. Je j'ai déposé, j'ai fait adopter un amendement 2018 au code du service national. Entraînant l'obligation de fournir aux élus des Français de l'étranger, une liste des postes organisant des JDC en 5 ans, aucune réponse. Il est vraiment indispensable aujourd'hui à l'heure où cela devient un enjeu d'influence de rétablir d'assurer la pérennité pérennité de ces JDC je rappellerai aussi que le ministère des Armées qu'il en soit félicitée avait pendant la période du. Covid-19 mise. Au point des formations. JBC par Internet. Malheureusement les Français de l'étranger n'ont même pas eu cette possibilité là alors je connais les difficultés de certains postes. D'où l'introduction de cette notion de circonstances exceptionnelles, mais c'est vraiment un enjeu très important. N'en déplaise à mes collègues de France. Compagnie chers collègues. Et monsieur le rapporteur. Avis de la commission. La présidente pour revenir à l'objet de l'amendement. C'est un avis favorable car effectivement il prend en compte les circonstances exceptionnelles. Merci monsieur le rapporteur. Madame la Ministre à vie du gouvernement. La JDC est obligatoire, vous le savez, pour les jeunes français à l'étranger là-dessus il y a pas de doute, c'est d'ailleurs l'article L 114 tiré 8 212, 16 et 212 17. Donc elle. Évidemment si je prends l'amendement telle qu'il est rédigé, il est satisfait puisque c'est obligatoire. Maintenant j'ai entendu la vie évidemment de de monsieur le rapporteur. Le président. Je vais mettre un avis de sagesse parce que. Parce que de toute façon, c'est obligatoire, donc il faut l'appliquer. Voilà. Merci madame la ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement.

le. Merci madame le ministre d'avoir dit que c'était obligatoire parce que c'est peut être obligatoire, mais ce n'est pas s'organiser, d'où l'importance de voter pour cet amendement. Merci. Merci pour cette précision, je mets donc aux voix l'amendement 189 qui a reçu un avis favorable de la commission une sagesse du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté. Nous avons à l'article 12, un amendement de 146. Madame la Ministre. de sa tombe de cet amendement et d'étendre le dispositif de réparation intégrale à l'ensemble des créances dans le fait générateur est survenue dans les 4 années précédant celle de la publication de la LPM donc la rédaction actuelle de l'article 12 permet une application immédiate de la réparation intégrale à des demandes en cours d'instruction et, par conséquent. Ah des faits générateurs antérieur à la promulgation de la loi. Mais cette rédaction est imparfaite, elle conduirait pour un dommage ayant eu lieu à une même date à une iniquité entre les militaires qui ont enclenché des démarches pour obtenir réparation. Et ce qui ne l'ont pas fait cet amendement vise donc à éviter cet écueil ainsi le militaire qui est éligible à la réparation intégrale pourra bénéficier de cette clause de rattrapage à condition que le fait générateur soit survenu dans les 4 années civiles précédant celle de la publication de la loi et donc c'est en cohérence avec la durée de la prescription quadriennal retenu par la loi du 31 décembre 1968. C'est un avis favorable. Madame la présidente. Parce que la mesure est favorable aux militants, aux militaires qui jusqu'à présent, s'était vu opposer un refus de réparation intégrale dans ce laps de temps. Avis favorable. Merci monsieur le rapporteur. Je mets donc aux voix l'amendement 246 du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission qui est pour. Qui compte qui s'abstient il est adopté, je mets aux voix l'article 12 qui. Pour qui compte. Qui s'abstient il est adopté après l'article 12, le 248. Madame la ministre. Merci madame la présidente. Donc, l'amendement a pour objet de clarifier et de rationaliser les critères d'attribution de la qualité du combattant et des avantages qui en constituent le corollaire. L'attribution de la qualité de combattants traduit la nécessité impérieuse pour la nation de reconnaître l'engagement de ceux qui ont assuré son salut en participant, soit à des conflits armés, soit des opérations. Ou des Ou des missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux en France. Face à la multiplication des opérations extérieures, il apparaît aujourd'hui nécessaire de clarifier et de rationaliser les conditions d'octroi de cette qualité. Cette reconnaissance s'exprime notamment par la délivrance de la carte du combattant délivrés en cas de participation à des actions de feu ou de combat ou après au moins 4 mois de service accompli sur un théâtre un théâtre d'opérations. Or, compte tenu des contingences matérielles liées aux conditions de rapatriement des troupes ce caractère fixé. Par la loi apparaît très rigide, il génère en pratique des inégalités au détriment de certains militaires. Contraint de quitter le théâtre juste avant d'avoir accompli cette durée de quatre mois. Ce sont ainsi 200 militaires par an qui se voient refuser la carte du combattant pour parfois moins d'une semaine de service en opérations extérieures, jusqu'à même juste un jour. Il s'agit d'une situation insatisfaisante pour y remédier au regard de la reconnaissance que la nation doit ces combattants. Il est donc prévu de renvoyer au pouvoir réglementaire, le soin de définir cette durée, cela permettra. Ainsi d'en assouplir les règles de computation en fixant cette durée à 16 semaines et en précisant que toute semaine commencer sera intégralement pris en compte cette situation ne modifie nullement le seuil de participation aux opérations extérieures aujourd'hui exigé à titre subsidiaire le présent amendement constitue également l'occasion de clarifier la rédaction imprécise des articles portant sur les conditions d'attribution de la qualité de combattants et de ses corollaires. Je souligne. Évidemment que c'est bien pour régler le problème de ceux auxquels il manque quelques jours voire même un jour donc abaisser légèrement le seuil et non pas bien sûr pour l'augmenter. Je crois que ça, ça il fallait le préciser. Et je suis bien évidemment dans une logique. Que de reconnaissance et non pas de rationnement. Donc je voudrais avoir aussi une pensée évidemment. Pour tous les soldats qui sont tombés en OPEX. Je crois que quand on travaille sur. Sur le le le la carte du combattant avec. Nos militaires. Je crois que ça c'est un amendement qui vaut d'être votée par toute l'assemblée. Merci. Merci madame la ministre, monsieur le rapporteur. le régime des combattants et celui des bénéficiaires de la reconnaissance de la nation, mais nous avions peur en lisant l'amendement que cette fixation par décret. Vise à augmenter la durée nécessaire pour bénéficier de ce statut, vous venez de dire que, au contraire, il s'agissait d'ajuster à la baisse la durée minimale et donc ça va dans le sens de l'intérêt de ces soldats et nous donnons un avis favorable. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. Amendement 247, madame la Ministre. Merci madame la présidente. Donc cet amendement a pour objet d'étendre l'attribution de la qualité de pupille de la nation aux enfants nés. Dans les 300 jours suivant le constat de l'incapacité de l'un des parents, c'est une attente forte des militaires et de leurs familles. C'est aussi une reconnaissance de leur engagement. l'extension de l'attribution de la qualité de pupille de nation aux enfants nés dans les 300 jours suivant le constat de l'incapacité d'un parent et non plus 300 jours suivant le rapatriement d'OPEX. Permettra une meilleure prise en compte dans le cadre de ce dispositif des aggravation d'affection et des blessures psychiques postérieur au retour en OPEX. Elle aura aussi le mérite de réduire les ruptures d'égalité dans les fratries en fonction de la date de naissance des enfants. Cette extension sera également appliquée aux enfants dans l'un des parents se trouve empêchée après avoir été victime d'un acte terroriste. C'est un avis favorable qui corrige effectivement une situation mais qui était parfaitement anormal puisque au sein d'une même fratrie un enfant pouvait être déclarée pupille tandis que sa soeur ou son frère ne l'était pas. Donc cela va dans le bon sens visant à la reconnaissance de l'État pupille de la nation, pour ses soldats. Qui. Ont Ont été soit blessés soit ont donné leur vie pour notre pays. Si monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement 247 du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il être adopté. Article 12 bis le 249. Fait du gouvernement Madame la Ministre on continue. Merci madame la présidente. Alors le le présent amendement. Est un amendement rédactionnel pour supprimer totalement le délai de carence de 90 jours en matière de présomption d'imputabilité des maladies en OPEX donc créé par un amendement gouvernemental, le numéro 11. Lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. L'article 12 bis du projet. De LPM supprime le principe d'un délai de carence de 90 jours s'agissant de la présomption d'imputabilité au service d'une maladie survenant en OPEX. L'évocation du délai de carence ainsi supprimés. Si. Subsiste toutefois dans un alinéa du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre le présent amendement purement rédactionnel vise à supprimer cette scories. Merci madame la ministre, monsieur le rapporteur. Avis favorable. Si je mets aux voix le 249 du gouvernement qui vient de recevoir un avis favorable. Qui est pour. Et contre. Sébastien, il est adopté. Je me vois l'article 12 bis. Qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient il est adopté. Article 13 je le mets aux voix même vote il est adopté. Après l'article 13 178. Monsieur Gontard le présente monsieur le président. Oui merci merci madame la présidente. Cet amendement vise à améliorer la protection des lanceuse et des lanceurs d'alerte dans l'armée afin de bien comprendre les enjeux, il faut remonter à 2002 1016 et plus précisément à la loi du 9 décembre 2016 qui a consacré un certain nombre de protection pour les lanceuses et lanceur d'alerte dans les entreprises privées, mais aussi dans l'armée. Cette loi était déjà une bonne avancée, mais la protection des lanceurs et lanceuses d'alerte restait toujours incomplète. Ces hommes et ces femmes s'expose à d'énormes risques et sont souvent victimes de représailles et que la. Rétrogradation l'intimidation de fichage. Dans ce contexte, une directive européenne de 2019 est venu compléter les protections déjà existantes. La loi du 21 mars 2022 a permis de transposer cette directive en droit français. En particulier, cette loi a permis de mieux protéger les personnes qui est d'une lanceuse ou un lanceur d'alerte. Il peut s'agir d'autres employé de l'entreprise ou encore des associations engagées pour la transparence qui savent ce que ce qu'il faut éviter et à qui il faut confier les informations. À cette occasion certaines de ces dispositions ont été élargis aux militaires plus spécifiquement un amendement de la rapporteure Madame Catherine Di Folco que je tiens à remercier a rendu les articles 6 8 11 12 hein et 13 applicable aux militaires. Mais à l'époque. Cet amendement a omis de rendre applicable militaires l'article 6. Or il s'agit pourtant d'un article essentiel parce qu'ils protègent les personnes et dans les danseuses et lanceur d'alerte cet amendement permettrait de corriger cette omission pour protéger les personnes physiques en lien avec les lances des lanceurs d'alerte ainsi que les facilitatrice et les facilitateurs merci. Oui madame la présidente. En réalité, cet amendement est satisfait par le dispositif qui a été évoqué par notre collègue. La loi du 21 mars 22 a en effet inséré dans son article 6 tirer hein. Relatives aux lanceurs d'alerte. Elle a ainsi romantique qui étend le dispositif de protection aux facilitateurs, ce qui est de bonne foi, les lanceurs d'alerte et cette extension vaut pour tous les cas de figure que le facilitateur soit salarié du privé, fonctionnaires ou militaires. Donc, je propose de retirer cet amendement. Puisqu'il est satisfait, sinon l'avis de la commission sera défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Oui mais présente en effet la loi avait déjà prévu d'intégrer comme la dit le le président Cambon. La loi avait déjà prévu de d'un d'intégrer cette affaire donc c'est déjà satisfait demande de retrait. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur Gontard vous le retirez vous le maintenez. Il est retiré. Je vous remercie donc le 178 et retiré. Nous passons au 179 rectifié. Merci madame la présidente. Seulement les actes répétés constituent du harcèlement, c'est la spécificité de cette infraction qui la rend à la fois difficile à poursuivent et aggravent encore la situation pour les victimes. Cependant la définition du harcèlement est beaucoup plus complexe, il peut arriver que la victime soit harcelée par plusieurs personnes qui se concertent. Dans ces cas, les actes de chaque auteur peuvent paraître isolé si les actes des autres auteurs ne sont pas prises en compte. Si tout le système qui est derrière et prudente compte il apparaît cependant que ces actes constituent bel et bien du harcèlement. extrêmement grave ces situations extrêmement graves sont restées méconnues jusqu'à ce que la loi du 2 août. 2021 pour renforcer la prévention de en santé au travail a enfin permis d'élargir la définition du harcèlement. Quant au harcèlement sexuel. La loi reconnaît désormais que des salariés subissant des propos de comportement venant de plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée peuvent également être victimes du harcèlement sexuel. Sauf que la loi de 2021 n'a modifié que le code du travail. Elle ne s'applique pas aux militaires, il est urgent d'y remédier et d'élargir la définition du harcèlement dans le code de la défense. De plus, cet amendement permettrait de reconnaître le harcèlement sexiste. Il est reconnu désormais dans le code du travail, mais toujours pas dans le code de la défense. Tout ce que nous proposons c'est de le c'est de le mettre à jour pour l'harmoniser avec le code du travail. Cette modification apportera une réelle avant une réelle avancée pour nos soldats car le harcèlement sexiste serait enfin reconnu la loi accorderait certaines protections aux victimes par exemple, le fait d'empêcher la victime de signaler un cas de harcèlement sexiste serait puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 euros. Merci. amendement qui vise à aligner la définition du harcèlement sexiste. Inscrit dans le code de la défense à celle beaucoup plus large et précise du code du travail est évidemment la bienvenue. Un avis très favorable. Merci, monsieur le Ministre, oui même avis, avis favorable. Si je mets donc aux voix le 179 rectifié qui a reçu 2 avis favorable. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. À un moment de en 180 rectifié. Monsieur Gontard le défend. d'un amendement de notre collègue Mélanie Vogel. De la même manière que l'amendement précédent cet amendement vise à mettre à jour le code de la défense pour tenir compte d'une évolution législative récemment intervenu ici il s'agit plus concrètement d'adapter la définition du harcèlement moral applicable aux militaires, d'une part il s'agit de définir le harcèlement moral comme agissements comme c'est actuellement le cas mais comme propos ou comportements terme utilisé par le code pénal, de l'autre par notre amendement permettrait de tenir compte des situations spécifiques du harcèlement exercé par plusieurs auteurs en mettant ainsi à jour la définition du harcèlement. Nous visons à mieux protéger nos militaires et à faciliter les signalements de ces faits, a-t-il d'exemple qu'il s'agirait d'interdire une suspension des militaires qui signalent des faits de harcèlement. Ces modifications peuvent paraître technique mais elles sont essentielles pour ces centaines de militaires qui sont victimes de harcèlement dans nos forces armées, tel est le cas par exemple d'Antoine, qui a témoigné dans l'émission complément d'enquête en juillet 2 villes, 22 au 1er jour avec son escadron d'une base aérienne encore si les cagoulés par ses nouveaux camarades qui attache ses mains ses chevilles avant de l'attacher à un poteau qui sert de cible pour des essais de tirs avec des avions de chasse ses camarades nous laisse là, immobile, il ne peut rien faire quand un avion de chasse tirent à balles réelles sur des cibles à proximité. Le bizutage, Antoine a été victime et tout simplement évidemment inacceptable mais, pire, il n'est pas la seule victime le bizutage et le harcèlement sont malheureusement systématique et trop souvent couverts par la hiérarchie militaire. Il faut des changements concrets et palpables notre amendement vise à apporter une brique à cet édifice en mettant à jour la définition du harcèlement moral dans l'armée. Merci. Les dispositifs et donc harmoniser cette définition du harcèlement moral dans le code de la défense, et cette fois-ci dans le code pénal. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. Alors évidemment sur le fond là aussi comme pour le moment précédent favorable on me signale juste. Une erreur dans le le fait de pointer. Dans la rédaction du code pénal sur le harcèlement moral, il y a deux de définition. Le harcèlement moral en général et le harcèlement moral au travail. Le législateur avait. Évidemment souhaité définir le cadre de ce qu'était le harcèlement moral dans le cadre du travail et donc au fond c'est une

en l'espèce pour permettre quand même d'avancer. Moi je vous propose un avis de sagesse. Sous-entendu favorable sur le fond mais quand même peut-être à charge législateur dans. Le le la CNPE ou les étapes suivantes, le cas échéant de peut-être reprendre la rédaction qui soit la plus efficiente, parce que vous savez que pour tout cela produisent leurs effets évidemment faut que la rédaction, soit la plus et puis les autres en tout cas le fond et là donc favorable. Merci monsieur le ministre, on a bien étant lu les remarques mais nous avons donc. Cet amendement 180 rectifié Monsieur Gontard Kémi. Aux voix avec un Aux voix avec un avis favorable de la commission. Si on est un une sagesse favorable, Monsieur le ministre, sous réserve de petits ajustements futurs en tout cas une sagesse favorable du gouvernement je le mets donc aux voix qui est pour. Qui compte qui s'abstient il est adopté après l'article 13 toujours le 288 du gouvernement, Monsieur le Ministre. Est nom du gouvernement mais il est aussi assez personnels. Ayant été confronté à un certain nombre de difficultés liées à des familles des conjointe ou conjoint de soldats tués. En mission dans lequel vous le savez on fait toujours une proposition particulière. Au conjoint survivant. S'il le souhaite, s'il le peut, si le besoin en est d'intégrer le ministère des Armées. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui le cadre d'emploi dans lequel nous pouvions proposer des choses étaient systématiquement dans les filières administratives. Or, pour tout un tas de cas pratiques très concrets sur lequel je ne rentrerai pas ici au fond on souhaite élargir à la capacité de le faire pour les catégories B. De la fonction publique, ce qui élargit le Champ du possible dans les unités ou dans les différents services du ministère dans lequel on peut proposer des choses donc c'est un amendement fondamentalement plein de blond Et qui permet évidemment de régler quelques cas bien précis. C'est. Merci monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. C'est une mesure effectivement pertinente qui va permettre à ces personnes déjà touchées par un malheur personnel important. De d'utiliser leurs compétences. Dans un ministère qui correspond plus à leur savoir-faire et à leur formation à vif. Sur le vif. Sur le rapporteur je mets aux voix le 288 avec un avis favorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté. À l'article 4. Plusieurs amendements 250 Monsieur le Ministre, amendement du gouvernement. Oui ma présence je je me battrai pas évidemment mais. Humaine ou naturelle. Pourquoi préciser ces 2 aspects si on on va là. On a oublié technologique, donc en fait on avait mis que le mot les menaces au pluriel. Comme ça. L'acceptabilité ou l'acceptation évidemment de la terminologie était globale là en précisant humaine ou naturelle. On en discute de facto beaucoup d'autres donc je, je viens vous proposez de réécrire comme ça l'été initialement dans la version sortie de l'Assemblée nationale tout simple. Merci monsieur le ministre, monsieur le rapport. Avis favorable. Très bien je me vois l'amendement 250 qui a reçu un avis favorable de la commission qui. Pour. Qui est contre. Qui ça. Tiens il est adopté le 114. Monsieur, Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de la ligne 12 de l'article de 14 traitant des droits à l'avancement des militaires d'active effectuant des activités dans la réserve opérationnelle à l'occasion de leur placement en congé pour convenances personnelles ou en congé parental porteuse d'une ambiguïté susceptibles de peau de conduire à une mauvaise interprétation du droit. Je m'explique cet alinéa du projet emploi en effet le terme de ses congés qui renvoie aux congés évoqué à La Linea actuel du code de la défense. Or, s'agissant du congé pour convenances personnelles ce cet article, l'article en question n'évoque que celui pris pour élever un enfant. Tandis que l'alinéa ajouté par la programme la présente LPM lui s'applique à tous les types de congé pour convenances personnelles et pas seulement à ce prix pour élever un enfant. Donc il est proposé, il vous est proposé. Mes chers collègues, de lever cette ambiguïté en énonçant explicitement à Lille l'alinéa 12 de l'article 14. La nature des congés visés. Merci. Oui ça va dans le bon sens évidemment. Donc, avis favorable, Monsieur le. Je mets aux voix l'amendement 114 qui a reçu 2 avis favorable à pied. Pour qui est contre. Il s'abstient il est adopté le 251 du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. En fait c'est aussi sous forme d'un moment d'appel et de et de questions. C'est pas un point dur, mais pourquoi avoir restreint le Champ des organismes. Le public dans lequel les réservistes peuvent servir la terminologie initial permettait au fond de les détacher. Dans toute forme de structures telles que on revient à la rédaction on les limites. Donc je sais pas quelle est l'intention du législateur qu'il a été poursuivi en commission. Voilà. Merci monsieur le rapporteur. Avis de la commission. En réalité la rédaction qui a été adopté en commission est conforme à la position qui a été prise par le Conseil d'État dans sa dans sa décision du 30 mars 2023 qui a proposé, je cite, de ne pas retenir la rédaction du du projet du gouvernement et le Conseil d'État recommande de lui substituer une mention des différentes catégories de personnes morales dans lesquelles cette affectation serait désormais possible. Ça veut donc dire qu'il y a une forme d'imprécisions dans la rédaction du gouvernement. C'est pour ça que la commission a émis un avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre, vous souhaitez la parole. Ben justement non puisque la rédaction de l'Assemblée nationale et celle du Conseil d'État. Donc la la rédaction ne fois plus s'il faut avancer en avance mais. C'est pour aussi montrer ma bonne foi comme je disais tout à l'heure au président Retailleau là on a la rédaction du Conseil d'État. le nombre d'établissements. Enfin le la série des établissements publics dans lesquels on peut détacher des réservistes. Donc je le dis là on apporte une rigidité et un cadre restrictif, là où on peut prendre des réservistes. Or, comme je vous connais bien et que je sais que, par ailleurs, ce n'est pas ce que vous souhaitez faire. Je m'interroge donc sur la rédaction en espèce d'où. Me permets d'insister sur cet amendement mais je sais que j'ai un succès limité quand j'insiste Dans son point 18, je lis le Conseil d'État considère en effet que le terme d'organismes n'a pas de contenu juridique, il est trop indéterminé et donc le Conseil propose de lui substituer la mention différentes catégories. Ce que j'ai dit tout à l'heure de voix. La décision du Conseil. vous mais j'ai pas les décisions du Conseil d'État à l'Assemblée nationale quand même. Si vous le voulez bien je vais donc mettre aux voix l'amendement 251 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 294. De la commission des Affaires étrangères, présenté par monsieur le rapporteur Cambon. Rédactionnelle. Ah ville favorable favorable du gouvernement sur l'amendement de la commission de 194. Qui est pour. Qui compte. Qui s'abstient il est adopté le 252 du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. Bon là je dois bien avouer que j'ai, j'ai besoin aussi de comprendre l'intention du législateur dans ce qui a été introduit en commission. Et c'est pour ça que nous proposons de le, de le supprimer, puisqu'en fait, là il s'agit de créer une obligation. Pour un réserviste opérationnel pas héros de mais héros hein, je précise bien. De rester disponible pour le ministère des Armées, 5 ans. Après que le contrat que l'engagement à servir dans la réserve soit tombé. Je ne vous cache pas que je je trouve la mesure. Au moins les clair mais elle est particulièrement brutal et dur. Puisque les réservistes opérationnels. Je ne parle pas de la héros de hein la disponibilité pour les anciens militaires on elle reviendra plus tard, c'est une autre affaire quand on est militaire d'active, on s'engage à des choses, c'est connu. Mais pour la R O un statut de réserviste opérationnel que vous connaissez bien. S'engager dans la réserve. Et avoir cette épée de Damoclès ou 5 ans après avoir quitté la réserve. Vous pouvez être rappelé de manière obligatoire. Quelle que soit parce que situation familiale. Quel que soit votre situation professionnelle est quelque chose qui me sont fondamentalement de parler dans le bon sens. Déjà parce que la Réserve doit rester un engagement de bon coeur, si j'ose dire sinon c'est tout notre modèle de réserve. Enfin c'est pas un service militaire, la réserve. c'est un engagement ont par définition ça suppose forcément l'adhésion. Du militaire de réserve. Que de, je pense qu'avec ce genre malheureusement de D'obligation c'est s'agit de ça hein. On dissuade beaucoup de gens à intégrer. La réserve opérationnelle. Et donc en fond, vous avez 20 ans vous décidez de signer un ESR et si vous le levez ou vous y mettez fin à 30 ans. En fait, on peut aller vous recherchez jusqu'à vos 35 ans. Alors je sais que j'ai peu de chance de faire adopter un amendement du gouvernement. Tout simplement parce que j'ai bien compris qu'il venait du gouvernement c'est pour susciter un peu la. La, la réalité c'est que là, j'invite véritablement le le législateur à faire preuve quand même de prudence parce que je trouve que la mesure est particulièrement brutale, moi j'aurais du mal à la défendre. Je vous le dis pas pour des raisons politiques hein mais en tant que réserviste moi même si on m'avait dit que j'avais cette obligation de rappel pendant 5 ans après la fin de mon ESR je ne suis pas certain que j'aurais signé cet si jeune. Donc là je je je vous demande véritablement de regarder si on est si un débat on peut après évidemment sous-amender enfin faire ce qu'il faut mais je pense que c'est un point clé. Et après on reprochera peut-être de dire des choses dans la presse mais là je crois vraiment qu'il faut prendre le temps quand même de légiférer dans le bon sens sur cette affaire. Merci monsieur le ministre, monsieur le rapporteur.

Cet amendement va plutôt dans le sens que vous souhaitez, puisque vous souhaitez. Accroître et mettent en oeuvre la montée en puissance des réserves opérationnelles de 1er et de 2ème niveau donc en offrant cette possibilité. Au contraire, on s'adresse à des réservistes qui choisissent et qui n'ont pas l'obligation. Il est pas question d'obliger qui que ce soit à commencer par vous et par mois. Qui en somme de. De continuer à être en disponibilité pendant 5 ans, donc je pense qu'il a peut-être une mauvaise perception. Du travail que nous avons voulu faire en commission. Donc si on maintient sa position, notre avis est défavorable à votre amendement. Quand. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup monsieur présent pour pour l'explication parce que de fait, je ne vois plus j'ai j'ai pas compris là le sens de la rédaction. Le problème c'est qu'en fait si c'est pas obligatoire. À quoi ça sert. Mais en quoi ce ça change de ce qui existe déjà. C'est ça que je ne comprends pas, parce que par définition. Le SR. On y reviendra sur les limites d'âge et cetera. La Commission modifier des choses qui me semble-t-il, vont dans le bon sens et autres mais en fait si c'est une option, c'est déjà largement couvert par ailleurs. Et dans la rédaction, je la lis juste le 1er complété par les mots et dans la limite de 5 ans à compter de la fin de leur engagement, sauf en cas de refus explicitement mentionnée par le réserviste. Alors vous êtes quand même en quelque chose, il va falloir que le réserviste quand il sera rappelé et un acte pour le refuser. 5 ans après. On est déjà dans un Champ on commence quelque chose qui comment cet le parcours de quelque chose d'obligatoire, qu'on le veuille ou non. Enfin je je lis hein, moi je ne fais plus je je je suis prêt à prendre toute forme de sous-amendements je sur les réserves. Je veux qu'on aboutisse à quelque chose de bien de fort donc mon propos n'est pas polémique, je le redis. Mais là vous avez quand même quelque chose ou droit dans la partie normatif de la LPM. Il est dit quand même que à réserver. 5 ans après avoir lâché son ESR devra quand même avoir un acte positif pour dire ah non explicitement. Je ne veux pas être appelés en cas de rappel. C'est le début du commencement de quelque chose qui a le parfum d'une forme d'obligation qui traîne par là ou alors c'est pas du tout obligatoire et vous l'avez dit alors de bonne foi je évidemment je crois bien volontiers, mais auquel cas qu'est-ce que ça change par rapport au cadre actuel. Donc en fait je moi par prudence je je vous le dis, ça évitera bien des confusions et des instrumentalisations aussi de par quelques milieux antimilitaristes qui pourront dire des choses divers et variés sur cette affaire. Moi je pense qu'il vaut mieux soit adopté l'amendement du gouvernement pour supprimer ce passage, ce peut être prendre le temps de sous-amendé pour mais laisser le texte en l'état ne me semble pas une bonne chose pour pour cette affaire, je dis vraiment de bonne foi. Madame Jourda, pardon, vous avez la parole pour explication de vote. Simplement apporter donc des précisions puisque il y a réservé réserve et il y a quelques années nous avions commis à la commission des Affaires étrangères en rapport avec Jean-Marie Bockel, qui était sur la Garde nationale. cet amendement vise particulièrement la partie Garde nationale qui ne, qui ne comprend pas dans ses réserves exclusivement donc Réservistes donc militaire mais qui comprend aussi des personnes donc de la police nationale. Donc le le. Le sens de cet amendement. C'est tout simplement en cas donc de menaces et singes une obligation bien parti. Puisqu'il y a possibilité c'est une ouverture en fait c'est que le réserviste qui voudra parce que donc ces conditions d'âge le lui permettent. Parce que c'est une catégorie de réservistes bien particulière. Faire un engagement supplémentaire, on le fera. Ce n'est pas une contrainte, c'est au contraire une ouverture et ça conforte ce que vous avez toujours souhaité que vous nous exprimer, c'est-à-dire le fait de faire remonter les effectifs et les réserves. Je ne vois pas où est la difficulté. Merci madame Jourda. Monsieur le Ministre.

Si vous voulez garder l'esprit de l'amendement. Moi je suggère une modification mais de taille quand même. C'est-à-dire celui qui termine son engagement dans la réserve, signale le fait qu'il veut rester dans une forme de réserve de la réserve mais par un acte positif après on racontera ce qu'on veut, on est en train de cuire dans la loi, on est en train de, de mettre en place une ficelle que l'on laisse au pied du réserviste pendant 5 ans. C'est factuel. Je si vous l'assumer collectivement telle quelle. On y va Dans les faits, je doute qu'en fait on l'assume complètement jusqu'au bout, je vous le dis comme je le pense et ça aura un effet à mon avis dissuasif sur les engagements dans la réserve. Donc on revient aussi ce que nous disions tout à l'heure sur l'économie générale du texte

Monsieur le rapporteur. Vous souhaitez la parole. Oui je. Fort des explications que vous donnez, je propose de préparer pour le. Dans le cas de la CMP un sous-amendement qui ira effectivement dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire l'inversion du dispositif. une c'est une très bonne chose. Retrait de l'amendement du gouvernement et réécriture dans ce, dans le sens que le présent comme on vient d'indiquer. Si Monsieur le ministre et donc l'amendement 252 et retiré. Le 253. Monsieur le Ministre, amendement du gouvernement. Pour le coup sur de défendu je rentre pas dans les détails. Je pense que sur une réserve opérationnelle héros de un mois c'est mieux que de moi, mais une fois plus, c'est pas un point un Monsieur le rapporteur. La commission donne un avis. Défavorable parce que diviser par 2 le préavis qui s'imposent aux employeurs d'anciens militaires est une charge supplémentaire pour eux donc on ne donne un avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. On le multiplie par 2, justement on ne le divise pas par deux, mais peu importe.

En tout cas je mets aux voix l'amendement 253 qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. S'appuyant il n'est pas adopté. 2 amendements identiques, faisant l'objet d'une discussion commune le 254 monsieur le ministre. Oui, coordination il est défendu et avis favorable à celui qui, celui du président comment.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, dans la lignée des des des articles traiter rapidement. Je vais essayer de de de de garder cette. Cette vitesse cet amendement propose d'ouvrir la possibilité notamment détendre les jours de d'autorisation d'absence par un accord entre l'employeur et l'employé accords devant être signé par les 2 parties et annexé au contrat de travail en effet au regard du rôle majeur qu'qui exerce aujourd'hui la réserve opérationnelle au sein de nos armées. Il s'agit de permettre aux femmes et aux hommes qui la composent, de s'investir davantage au service de la France, cette mesure leur permettra d'aller au-delà du minimum prévu par la loi. Dans l'hypothèse où leur emploi le permet bien évidemment et que leur employeur il consent. Merci Monsieur et monsieur le rapporteur. Alors cet amendement. La présidente et tout à fait en cohérence avec l'assouplissement du régime soutenu par la Commission, donc nous donnons un avis favorable. Merci. Monsieur le Ministre. Oui a priori ils seraient déjà satisfait par la loi des partis, mais bon, le cas échéant si doutes ça. Allez. Le 168 reçoit donc un avis favorable de la commission et une sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. 291 du gouvernement défendu et défendu. Favorable. Je mets aux voix le 280 du gouvernement avec un avis favorable qui pour qui est contre qui s'abstient il est adopté. Je mets aux voix l'article 14 qui est pour qui est compte qui s'abstient il est adopté. Ah d'accord. Ensuite. Près l'article 14, le 9 rectifier bis monsieur Lévy le défend. merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur et le président de la commission. Mes chers collègues, la réserve citoyenne créée par la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du Service de défense constitue une initiative louable qui renforce les Liens entre civils et militaires. En effet, le réserviste citoyen, en tant que collaborateur occasionnel du service public contribue efficacement au service des forces armées. Il existe de nombreuses réussites dans ce domaine. Bien que leur nature varie en fonction des régiments certains réservistes citoyens ont l'opportunité d'accomplir des missions particulièrement intéressante pour le régime en détachement. C'est le cas dans mon département, que ce soit la base de Défense ou au 17ème régiment du génie parachutiste cependant dans d'autres cas certains réserves citoyens peuvent avoir l'impression de ne pas être utilisées à leur plein potentiel et peut finalement se sentir en marge de leur régiment. Cet amendement vise à renforcer le sentiment d'appartenance des réserves et citoyens aux forces armées, en leur permettant de porter un uniforme ou un signe distinctif, lorsqu'ils sont en service. Il s'agit d'une mesure volontaire qui ne vise pas confondre les réservistes citoyen avec les réservistes opérationnels mais plutôt à renforcer leur engagement et leur identification à l'armée. Cette mesure pourrait également faciliter la reconnaissance des réservistes citoyen lors de leurs interventions en cas de besoin extrême. Je tiens à préciser que j'avais déposé également 2 autres amendements portant sur la réserve citoyenne qui ont malheureusement été rude déclarée recevable le 1er vise proposer sur la base du volontariat. Une formation militaire basique aux réserviste citoyen et le second vise à fournir une carte d'identité militaire avec la mention réservé citoyen comme c'est le cas dans la gendarmerie nationale. Le 1er été déclarée recevable otite de l'article 40 second au titre de l'article 41. Pas de chance, cependant Monsieur le Ministre, je pense que ce débat mérite d'être ouvert, je vous remercie. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Avis de la commission. Je donne un avis favorable sur cet amendement, car je crois que la possibilité pour. Un membre de la réserve citoyenne de défense de porter l'uniforme qui été confiée ou le signe distinctif. Est un élément important pour. Donner un rôle évidemment évidemment qu'il soit cadré lors des manifestations mémorielles par exemple. Il s'agit pas de porter cet uniforme dans n'importe quelle circonstance, mais je crois que ça peut être une bonne chose et au moins l'insigne, je vous remercie. Avis favorable. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. Alors là aussi le diable se niche dans les détails parce que. Un uniforme ou un signe distinctif c'est 2 choses différentes. Donc le signe distinctif pour être honnête avec vous, j'y suis favorable. L'uniforme. J'y suis défavorable puisque, porté l'uniforme c'est être militaire. En tout cas dans les forces armées, soit vous êtes militaires d'active et vous portez uniforme vous êtes militaire de réserve opérationnelle et vous êtes convoqué et vous portez l'uniforme. Vous êtes réservé citoyen. C'est ainsi que les doctrines ont été imaginées. Vous n'êtes pas militaire. Donc moi je peux te favorable à cet amendement. Si on enlève le mot uniforme sur signe distinctif. Aucun problème, il existe d'ailleurs faut sûrement qu'on réfléchisse à améliorer tout ça et des réflexions aussi à mon avis à avoir sur les grades. Moi j'ai beaucoup de retour aussi dans les forces armées où il a parfois un peu de confusion, il y a des lieutenant-colonel les colonels les capitaines de vaisseau dans tous les sens. On fera sûrement réfléchir aussi un tout petit peu à tout ça. Néanmoins, j'insiste. Sur le fait que quand on porte l'uniforme c'est que on a une légitimité pour le faire et la légitimité, c'est qu'on est militaire a réservé citoyens tels que ça fonctionne n'est pas militaire, donc si vous en êtes d'accord. Avis favorable si vous rectifier l'amendement en enlevant le mot uniforme et ont bel et on pour le le signe distinctif. Après si il n'y a pas de modification de l'amendement, avis défavorable, pardon du caractère binaire. Mais je pense que le port de l'uniforme dit quelque chose dans les forces armées tout ça les et ceux qui les connaissent, vous en savez quelque chose et qu'on ne peut pas banaliser ce cette affaire c'est comme le port de l'écharpe pour le maire ou le maire adjoint, le conseiller municipal peut le porter dans des conditions spécifiques lorsqu'il Marie par délégation du maire et tous ces symboles ont. Ont toujours une histoire dans notre République et donc je pense qu'il faut, il faut qu'on fasse attention à, à bien ne pas trop s'éloigner de l'histoire et les traditions de nos armées le cas échéant. Merci, monsieur le Ministre, alors. Monsieur le rapporteur. D'abord, puis monsieur Perrin, puis Monsieur Guerriau. L'insigne ne ressemblent pas à un insigne de supermarché fait quelque chose de digne, pour que ces réservistes qui participent à notre vie locale soit effectivement l'objet d'une distinction particulière. monsieur le rapporteur. Alors d'abord Monsieur Lévy puisque monsieur Lévy a demandé la parole et ce serait bien de savoir d'abord quelle est la position de monsieur Lévy sur la proposition du ministre avant de laisser les explications de vote s'exprimer. Alors Monsieur Lévy. Dites-nous si vous êtes d'accord sur les propositions, pas de Monsieur le Ministre.

Un uniforme ou une tenue. Vous pouvez l'apporter peut-être l'appeler différemment mais une tenue qui vient différencier ces réservistes à mon avis il est attendu et pour en avoir discuté avec également des chefs de corps. C'est une idée que leur paraît intéressante. Alors on peut peut-être le voter en l'état et ensuite y réfléchir

Les réserviste de la marine. Était en capacité de porter l'uniforme sur certaines cérémonies. Je crois que ça n'est plus le cas, mais que ce qu'il le faire continue quand même à le faire. Je porte pas de jugement sur l'uniforme, mais moi ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il est nécessaire et voir urgent. De créer les conditions pour que les réservistes citoyen soit reconnu. Je suis moi-même réserviste citoyen dans une régiment d'artillerie. J'ai quelques amis quelques collègues qui en font partie À l'heure où on voudrait développer davantage la réserve la réserve citoyenne est une réserve qui êtes importante parce qu'elle permet aussi un certain nombre de services dans nos régiments. Que ce soit des accompagnements dans diverses. Sur diverses modules de management et autres par différents chefs d'entreprise, en tout cas il y a une nécessité absolue maintenant de valoriser l'action des réserves citoyens qui aujourd'hui ne sont absolument pas reconnus en dehors d'un pin's qui dans l'armée de l'air et Éric effectivement relativement. Portable on va dire ça comme ça mais qui est dans l'armée de terre par exemple ressemble effectivement plus. Enfin, il est extrêmement lourd côté du côté où il est porté. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour valoriser cette action pour faire en sorte aussi que dans les régiments du chef de corps. Leur portes aussi davantage d'attention parce qu'on se rend compte aussi qu'ils sont très peu sollicité. Moi ce que je voudrais juste dire c'est que au travers de cet amendement de monsieur Lévy. Je pense qu'il y a aussi peut-être un appel à faire en sorte que les réserves citoyens soient davantage associés davantage. soit davantage mis en avant parce que c'était évidemment un geste, un geste qui n'est pas neutre que de s'engager comme réserviste citoyen il en faut davantage et peut être que ça peut aussi ouvrir des portes et offrir des services à nos armées, donc moi j'insiste sur le fait de la nécessité de les valoriser. Merci. Merci monsieur Perrin. La parole est à monsieur Merci madame la présidente. Mais moi je soutiendrai la proposition de notre collègue Lévy. D'abord parce que comme ça a été rappelé d'abord dans la marine nationale ont porté l'uniforme dans la réserve citoyenne, on le porter avec utilité puisque il y a des stages militaire qui sont organisées, auquel participent les réserves citoyen on peut considérer d'ailleurs que ça allait à l'issue de ces stages qui pourrait porter l'uniforme. D'autre part le problème de la marine nationale, c'est qu'elle est présente dans certains secteurs Hugard sa spécificité maritime et donc, dans beaucoup d'endroits, elle n'est pas présente. Donc c'est une représentation par l'uniforme sur les commémorations à un certain sens de représentation à proprement parler de la marine, puis enfin la notion d'uniforme, c'est pas seulement l'aspect militaire combien porte l'uniforme dans d'autres domaines. On a parlé du SNU tout à l'heure en disant que ce n'était pas lié à à la LPM et je partage mais pour autant il y a un uniforme pour le SNU. Donc je ne crois pas qu'on puisse relever l'idée que en aucune manière ont pu avoir ces distinctions par l'uniforme d'appartenir à une corporation quelle qu'soit que ce soit la réserve citoyenne, que ce soit les pompiers que ce soir des secouristes, que ça soit peu importe mais je pense qu'il y a une distinction en la matière qui peut être utile et puis encore une fois la réserve citoyenne, c'est quelque chose de très différent d'un corps d'armée à l'autre dans certains corps Alain une utilité plus forte que dans d'autres et puis l'initiative peut être de nature à faire en sorte que ah soit toujours plus utile avec les compétences qui sont relevés de ceux qui s'engagent dans réserve citoyenne. Donc moi je suis frais favorable à la proposition qui a été faite par notre collègue Lévy et donc je voterai dans ce sens. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Folliot. Oui merci madame la présidente, moi je comprends Monsieur le Ministre, ce que vous venez de dire et vos propos par rapport à la notion de tenue de de de de l'uniforme, mais aussi je partage tout à fait les préoccupations de notre collègue Lévy par rapport au fait d'avoir un signe réellement distinctif. À titre personnel, j'ai, j'ai l'honneur de servir comme réserviste citoyen auprès de la 11ème brigade de parachutistes. Mais au-delà du du du fait d'avoir une pince comme certaines d'entre vous l'ont et qui effectivement ne n'est pas très visible. Je me demande si une solution ne serait pas. Un compromis avec une forme d'écharpe. Que pourrait avoir et porté dans certaines circonstances, donc les réservistes citoyens qui permettrait de les Z'identifier visuellement, de pouvoir aussi leur permettre de pouvoir jouer leur rôle parce que c'est un rôle d'influence et comme vous l'avez dit, monsieur le Ministre il ne, à la différence de la réserve opérationnelle ou les réservistes donc joue un rôle très actif. Là c'est pas un rôle opérationnel mais c'est un rôle d'influence qui a son importance surtout. À un moment où. Le lien armée nation a tendance à se distendre à à certains égards, et donc je pense que tout ce qui permettrait de pouvoir faire de telle sorte qu'il puisse y avoir cette meilleure et Bourne reconnaissance donc des réservistes citoyen. Pourrait être un élément et une avancée tout à fait positive et significative. Donc essayons on peut être de voter cet amendement de tels quels et puis peut être Monsieur le Ministre, au moment de la commission mixte paritaire d'essayer de trouver un compromis qui permet de réaliser finalement quelque chose et qui permettent d'équilibrer le tout et et de pouvoir reconnaître donc le rôle de cette réserve citoyenne mais aussi de pouvoir respecter la différenciation entre réserve citoyenne et réserve opérationnelle au niveau de l'uniforme. Si cher collègue, la parole est à monsieur Alizart. Les ministre. Oui madame la présidente. Moi personnellement je fais partie de la réserve citoyenne de la gendarmerie depuis 2009. Je porte pas d'uniforme et ça ne me pose pas de problème particulier. C'est le 1er point le le 2ème point. Je crois qu'effectivement et ça a été dit par quelques collègues. L'activité des réserves citoyennes est extrêmement hétérogène d'une arme à l'autre et je dirais même d'un régiment ou. D'un rattachement à l'autre. Je connais des réservistes de la marine qui font effectivement des exercices des formations, des réunions régulières. Dans la gendarmerie en fonction du chef de corps que nous avions. Il était en poste 2 ou 3 ans il voulait nous faire travailler ont travaillé 2 ou 3 ans. Son successeur arriver il n'en voyait pas l'utilité et pendant 2 ou 3 ans on ne se rencontraient pas donc Monsieur le Ministre, un 1er point, peut-être qu'il faudrait veiller à donner une certaine homogénéité à cette fonction de la réserve citoyenne et sur la problématique du signe distinctif, je crois qu'effectivement le le pin's puisque c'est le terme qui a été adopté et peut être un peu faible, il y a peut-être une une solution intermédiaire a trouvé je livre ça à votre réflexion la réserve citoyenne de l'armée de terre rattaché au DM des du Calvados. Ils se sont mis d'accord sur un dress code. Ce n'est donc pas un uniforme mais ils ont tous le même pantalon, ils sont tous le même blazer une chemise de la même couleur et une cravate de la même couleur, avec ce fameux pince et je peux vous dire que quand ils sont ensemble dans une cérémonie ça de l'allure. On les reconnaît. Et ce n'est pas un uniforme. Certains portent le béret. Mais pour ce qui était dans les parachutistes avant parce qu'il se trouve aussi qu'on retrouve dans la citoyenne quelques anciens de l'active. Voilà c'est une suggestion. Mais je peux vous dire que ça fonctionne et on les reconnaît bien et il y a pas de confusion avec l'uniforme et je termine là- dessus. Le sujet de l'uniforme vis-à-vis des militaires d'active, ça peut être aussi un sujet. Si cher collègue, Monsieur le Ministre, vous avez demandé la parole. Ensuite on continue. Les explications de vote. Merci beaucoup présente un débat aussi passionné que pour les marges frictionnel. Donc ce qui m'amène à. à dire plusieurs choses hein. Oui il y a un sujet de, d'animation du réseau de la réserve citoyenne, il y a pas d'août Clairement. Identifié. Que. Comme l'a dit très justement le sénateur à Lisa ça va comme c'est mené ça dépend beaucoup de la manière dont les chefs de corps ou comment le groupement de gendarmerie. Le Maine et ça c'est quelque chose que j'ai bien bien en et qui d'ailleurs objectivement peut aussi concerner la réserve opérationnelle, puisque, on y reviendra sans doute peut-être dans d'autres cas de mais le degré de convocation des réservistes parfois dépend aussi du commandement et donc là moi j'ai toute une manoeuvre interne aussi importante avec les DNA et avec les gouverneurs militaires préfets maritimes et pour, évidemment. Faire en sorte que tout ça se donner 1er point. 2ème point parce que à force de renvoyer tout à la CMP au bout d'un moment je je vois aussi comment ça va se terminer, je vous propose un sous-amendement. Donc je suis amende en séance. Les réserves citoyen lorsqu'ils sont en service peuvent porter un signe distinctif donc mon sous-amendement sous un monde de suppression pour un uniforme. Conformément aux règles et régulations établi par le ministère de la Défense point cet insigne distinctif permet d'identifier clairement j'enlève uniforme.

On peut faire une commission ad hoc. Je peux vous soumettre les choses avant. Non mais je suis, je veux dire c'est pas un sujet blocage. C'est pas un sujet de blocage. En revanche je je trace la ligne quand même sur le mot uniforme. C'est-à-dire que il y a se différencier je. De fait, j'ai vu Monsieur le Sénateur Alizart et pour les cérémonies du débarquement et dans le petit village de meuble dans lequel j'ai quelques attaches comme vous le savez, j'ai vu nos amis citoyen dans une tenue distinctive. Mais vous êtes dans une loi de programmation militaire le mot uniforme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand vous êtes colonel de gendarmerie de réserves comme le sénateur Alizart. Ça veut donc dire que vous pouvez arriver avec un uniforme de colonel de gendarmerie d'active. Une cérémonie. Au passage, pour avoir. Moi-même été réservistes opérationnels pour le coup dans la gendarmerie. Vous faites quoi vous armer le sénateur Alizart pour sa légitime défense parce que quand on a marqué. Ça ne veut pas. Nommé. Pardon de poser la question mais il est temps. S'il a marqué gendarmerie sur son uniforme, vous ferez comment pour expliquer à nos autres concitoyens en fait qui n'est pas vraiment gendarmes d'active ou pas vraiment gendarmes opérationnel. L'uniforme veut dire quelque chose. L'uniforme n'est pas un déguisement je je le dis vraiment avec gravité et là je veux je suis aussi les responsables de 260 de 200.000 militaires qui n'ont pas envie de, de se confronter à des gens qui, même si ce sont des gens formidables parce que réserviste citoyen ne sont pas militaire. je je, vraiment, j'insiste et je pense que les sénateurs membres de la commission de la défense qui passe du temps avec les forces armées, vous voyez très bien de quoi il s'agit et monsieur le sénateur Perrin si les marins ne sont plus autorisés à le faire, c'est-à-dire pas sur une décision ministérielle mais sur une décision des chefs d'état major. C'est bien qu'il a eu des raisons. Des dérives. Avec de graves problèmes et donc. Il faut faire attention à ça. Et dernier point. Si on confond réserve citoyenne et réserve opérationnelle on va forcément tu es une des deux à la fin, c'est inévitable. Ce ne sont pas les mêmes missions. Le réserviste citoyen à des tâches d'influence qu'on peut sûrement mieux codifier c'est du réglementaire, donc ça si vous voulez qu'on travaille tous ensemble, moi je suis prêt, a précisé tout ce que vous voulez, il y a un cadre d'emploi on peut le faire évoluer, tout ce que vous voulez. Néanmoins, le réserviste opérationnel lorsqu'il est convoqué, il devient pleinement militaire si vous êtes colonel dans la réserve opérationnelle gendarmerie le jour où vous êtes convoqués, vous êtes militaire et vous avez tous les attributs tous les droits. Tous les devoirs. La solde et la discipline qui va avec. D'un colonel de gendarmerie là pour un site un une réserve citoyenne, vous êtes dans une zone dans laquelle vous restez civils donc en fait ça n'a l'air de rien, et ça paraît sympathique comme ça, au détour d'une phrase M. à 11h et Mais en fait on bascule dans quelque chose qui est très observée par les forces armées. C'est pour ça que je me permets d'être particulièrement. Lourd sur le sujet d'moins pour avancer et ne pas rester sur quelque chose qui serait mal écrit ou autre. Je vous propose ce sous-amendement qui permet de m'engager à faire évoluer tout ce que vous souhaitez sur la réserve citoyenne mais il y a pas le mot uniforme et croyez-moi, ça a du prix que de d'apporter ces clarifications. Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous repréciser pour la bonne rédaction du texte qui peuvent porter un signe ou un, un signe distinctif. Bah vaut mieux mettre signe comme ça ça laissera plus de place à l'interprétation de ce que vous voulez, ça peut te. Ce que vous voulez mais pas d'uniforme. Encore donc signe distinctif, je reprends la phrase les réservistes citoyen lorsqu'ils sont en service peuvent porter un signe distinctif conformément aux règles et régulations établi par le ministère de la Défense ce signe distinctif permet d'identifier clairement les réserver ce citoyen c'est ça. Exactement et donc le conformément aux règles et régulations établi par le ministère de la Défense. Je le mettrai en concertation avec vous à prendre avant de prendre le cas échéant une mesure réglementaire, voilà comme ça on est complet. OK. On reprend les explications de vote avant de mettre aux voix, cette proposition de sous-amendements et puis surtout on va demander à monsieur Lévy. Aussi son point de vue. Mais d'abord on finisse. Explications de vote comme ça. Allez. Madame Sollogoub.

Est-ce que il serait pas possible d'amender en disant qu'on porte une tenue distinctive, moi je partage complètement votre analyse sur le mot uniforme qui sera de toute manière mal perçu blessant. Ça peut être. Source de confusion. Mais ce que disait notre collègue Alizart a quand même du sens aussi Quentin un groupe porte la même tenue. Ça a de l'allure. On a l'impression d'appartenir encore. Les jeunes du service national universel, c'est tout simple. Ils ont le petit t-shirt le même pantalon, ça peut être quelque chose de simple. Les sapeurs-pompiers volontaires, les jeunes les JSP, bon on peut avoir une tenue similaire. Ça peut une tenue distinctive qui soit pas un uniforme c'était juste de la sémantique, je je suis d'accord avec vous pour uniforme mais ça peut être une tenue distinctive. Oui merci madame la présidente prend pas souvent le la parole dans cet hémicycle mais là franchement. Parler de de tenue. D'uniforme, c'est quand même une sacrée différence. Nous ne sommes pas des militaires.

Voilà, là dessus, je crois qu'on est peut-être plusieurs et d'accord et et je crois que c'est important. Alors maintenant qu'on est un signe distinctif, pourquoi pas mais ce qui est important là dedans, c'est notre engagement qu'on a c'est ça qui est important et j'ai pas besoin d'avoir un uniforme même. Même si j'en ai un. Pour me dire que je m'engage. Aux côtés par exemple du SMV service militaire volontaire. Et puis moi ce qui m'ennuie encore plus là-dedans, c'est quand on nous donne. Moi les grades. Moi les grades. C'est pour les militaires parce qu'ils ont passé des concours, ils ont passé tout un tas d'examens. Ils ont été au combat. Et grâce à ça, ils ont obtenu des grades et nous des fois on se retrouve lieutenant-colonel. Simplement parce qu'on a travaillé aux côtés du SMV ou je ne sais trop quoi, et parfois certains sont lieutenant colonel sans avoir rien fait. Hé ben ça ça me dérange encore plus. Voilà donc moi je ne voudrais pas en tous les cas, cet amendement pour tout cela, et et par contre oui peut être réfléchir pour qu'on ait peut-être une meilleure reconnaissance parce que je pense que c'est ça aussi une meilleure reconnaissance sur le terrain et qu'on ait une meilleure connaissance quand on est présent en tous les cas au niveau de des cérémonies. Voilà je vous remercie. Si beaucoup, je suis certainement le plus ancien dans la réserve citoyenne d'entre vous, puisque j'y suis entré dès la création, je venais de terminer Liège DN. Et je dois dire que j'ai quand même été aussi assez choqué de rentrer immédiatement au grade de commandant maintenant bien sûr tous les sénateurs, peut-être que le Neil mais je crois que c'est un vrai problème de fond parce que très honnêtement vis-à-vis des militaires d'active, j'étais gêné et je rejoins d'ailleurs ce que vient de dire ma collègue. Guinness. Mais comment en en arrivant juste OK avec l'IHD admet, certains n'ont même pas fait l'IHU ADN n'ont même pas de connaissance des enjeux militaires et ont immédiatement un grade de haut niveau et je trouve que c'est presque insultant pour des militaires d'active qui prennent le risque au quotidien qui peuvent donner leur sang, qui ont des responsabilités énormes et c'est vrai que j'estime mes chers collègues, que si nous sommes quasiment tous maintenant, colonel de réserve citoyenne dans différentes armes, nous devons l'être avant tout pour servir pour servir nos armées pour servir la France. Hé bien évidemment pas pour demander des avantages honnêtement cette question d'uniforme. Moi aussi ça me gêne qui est peut être un signe distinctif bien sûr pourquoi pas mais ce qui est important c'est de faire connaître la réserve citoyenne et surtout de la faire mieux accepter parce que je crois qu'il serait très important, Monsieur le Ministre d'entamer une véritable réflexion sur ce qu'est la réserve citoyenne, ça fait des années que je le demande, mais je n'y suis jamais arrivé mais ça me paraît important pour définir vraiment l'émission et l'encourager. Hé bien insister sur cette question de service parce qu'effectivement, je connais beaucoup de réservistes citoyen à qui on ne demande strictement rien, et ça je trouve que c'est très dommage. Merci. Je vous propose quand même de vous lire la proposition de sous-amendements. De. Du gouvernement il est en cours de distribution normalement vous l'avez vous

Et dans la seconde phrase remplacer les mots cet uniforme ou par le mot ce voilà. Ce qui est dans ce sous-amendement. S'il y a des explications de vote. d'abord, avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Sur ce sous-amendement. assez paradoxal de passer plus de temps sur cette affaire que sur la dissuasion nucléaire. Mais ce que je veux néanmoins dire c'est que derrière cette affaire d'uniformes et de si il y a la condition et la considération que l'on doit porter à la réserve citoyenne. Alors ça peut être une tenue. Ça peut être un signe. Tout ce que vous voulez mais moi qui assiste beaucoup à des prises d'armes à des prises d'armes des manifestations patriotiques. Je vois trop souvent des gens qui font partie de la réserve citoyenne et qui se plaignent de ne pas être traités comme il pourrait l'être alors que ce sont des personnes qui ont fait manifestement oeuvre de dévouement, par rapport à la cause militaire. Donc je vous laisse évidemment trouver le moyen nécessaire pour les distinguer. Merci. Avis favorable au sous-amendement. Non je voulais simplement madame la présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur rapporteur dire que je vais retirer mon amendement au profit du sous-amendements mais à qu'on y par contre. Non, non Monsieur Lévy vous retirez pas votre amendement en fait tiens. Ah d'accord mais il y a plus de sous-amendements. Alors parce que je voulais dire simplement c'est que on a parlé beaucoup de la gendarmerie, on a parlé beaucoup de la gendarmerie dans la gendarmerie. Vous avez une carte d'identité.

Notre signification effectivement donc je comprends vos remarques. Et j'accepte. J'accepte les modifications du sous-amendement. Alors donc je vais, si vous le voulez bien avec l'avis favorable de la commission mettre aux voix le sous-amendement. 310 proposée par le gouvernement. Donc avec son avis favorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Et je mets donc aux voix l'amendement 9 rectifier bis ainsi sous-amendé donc. Qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient il est adopté. Monsieur le ministre, acceptez-vous de faire sauter le gage de cet amendement. Je le crois oui. Si Monsieur le Ministre. Alors, nous passons un. L'amendement 122, il n'est pas défendu. Donc il tombeur. Et nous passons au 296. Monsieur le rapporteur. Rédactionnelle. Avis du gouvernement. Je mets aux voix le 296 avec son avis favorable qui est pour qui compte qui s'abstient il est adopté. Je mets aux voix l'article 14 bis qui est pour. Contre, abstention. Oui il est adopté, article 15 297. Monsieur le rapporteur. cet amendement vise à étendre les l'éligibilité au réengagement sous statut militaire aux anciens militaires qui ont bénéficié d'un congé de reconversion ou d'un congé pour création ou reprise d'entreprise. Merci Monsieur le Ministre, Plutôt avis défavorable, enfin. Sans qu'il ne soit tranchée. C'est juste que s'il y a eu un plan de départs déjà enfin une accompagnement pardonnez-moi vous créez quand même un effet trappe. Malgré tout, voilà donc je je les services du ministère redoute plutôt. Un effet pervers potentiels donc avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre, je vais donc mettre aux voix l'amendement 297 de la commission. Qui a reçu en David défavorable du gouvernement. C'est pour. Qui est contre. Qui s'abstient il est adopté le 205. Présenté par le gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui merci beaucoup amendement d'appel pour comprendre ce que vous souhaitiez faire. En commission. Excluant les volontaires de la réserve personnelle du dispositif de maintien au service de la limite d'âge en fait vous avez pris déjà une série de mesures qui me semble bonne, vous avez toutes. Sur une limite d'âge de 72 ans. Très bien. En commission, c'est ce que vous avez fait et je trouve ça très bien. Pour être honnête, c'est simple, c'est clair. Avec cette mesure là ça nous emmène jusqu'à 75 ans. Alors du point de vue des armées il y a pas de besoins en ressources humaines identifiées en tant que telle. Donc c'était juste pour comprendre ce que vous avez souhaité faire en commission. Je ne sais pas qui sont les auteurs de cet amendement en commission. Mais c'est pour comprendre. Monsieur le rapporteur. Le ministre, il s'agissait de maintenir en service pendant une durée maximale de trois ans des réservistes opérationnels, qui ont une compétence particulièrement recherché de de de la limite et qui pourrait bénéficier à la fois aux armées et aux réservistes qui en font la demande toujours le même principe du volontariat. Il y a pas de raison cachée, c'est franchement pour vous aider justement à monter en puissance sur le plan de la réserve. ça nous emmène à 75 ans mais j'ai rien contre hein. Donc. Si. Je le retire. Merci, monsieur le Ministre donc l'amendement 255 et retiré je mets aux voix l'article 15. Qui est pour. Compte. Abstention il est adopté. Article 16 même vote il est adopté. Article 1766 rectifié Monsieur Guillaume. Merci madame la présidente. L'article 17, créer le régime d'apprentissage militaire c'est une école, c'est une bonne chose pour à la fois susciter des vocations et raffermir le lien entre l'armée et sa jeunesse 3 établissements d'enseignement technique préparatoire militaires sont visés par ce nouveau régime. Pour l'armée de terre, il s'agit de l'école militaire préparatoire technique de Bourges pour la marine nationale, c'est l'école des mousses et enfin pour les, l'armée de l'air et de l'espace, c'est l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace. Il est tout à fait justifié à travers ses articles d'encadrer le temps de service des militaires mineurs conformément à nos valeurs et nos engagements conventionnels internationaux sur l'emploi des mineurs. Toutefois en harmonisant le statut des élèves des écoles techniques préparatoires militaire est un certain que cet article préserve les spécificités des 3 écoles que je viens de mentionner, chacune d'entre elles ont un effet des spécificités qui touche à l'âge aux conditions d'accès à la durée des formations et un désengagement proposés au terme de la formation au régime de soldes ou des permissions cet amendement vise à garantir le maintien de ses particularités. À chaque filière de formation d'apprentissage militaire dans la perspective des futurs décrets. madame la présidente. Si le Ministre s'engage à maintenir toutes ses spécificités. Je pense que cet amendement du reste devrait plutôt trouver sa place dans le rapport annexé au projet de loi, c'est pour ça que je propose le retrait. dans la suite du du rapporteur président il y a pas de volonté de bouger quoi que ce soit donc demande de retrait et le cas échéant. Merci monsieur Guy l'amendement 166 et retiré je mets aux voix l'article 17 qui et pour qui compte qui s'abstient il est adopté. Article 17 bis même vote, s'il est adopté. Je passe au 161 rectifié ce monsieur viol toujours. Notre collègue rapporteur et président de la commission, a rappelé le travail récent du Sénat sur la jeunesse et la citoyenneté qui a donné lieu l'année dernière à un rapport cet amendement est issu d'une des préconisations de la mission d'information d'anciens volontaires à l'insertion peuvent rencontrer des difficultés d'accès au logement et à leurs débuts dans la vie professionnelle. Un dispositif du code du service national propose à ces jeunes un contrat de soutien de 3 mois afin de leur permettre de continuer à être hébergés à l'Epide, établissement d'insertion dans l'emploi. Alors qu'ils ne sont plus volontaire à l'insertion, la durée de ce contrat qui constitue un outil non négligeable d'accompagnement au logement et mérite d'être étendue. Il s'agit de prolonger de 3 mois. Ce contrat de soutien. Ce qui le porterait à six mois maximum afin de ne pas créer une charge publique, il est prévu que cette faculté dépendent de logements existants disponible au sein de l'Epide je vous remercie. Oui alors avis défavorable pour une simple et bonne raison c'est que ce n'est pas le ministre de l'armée qui est mise tutelle des des épis mais ministère du Travail, donc. Non. Alors je mets aux voix l'amendement 161 rectifié qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement. Qui est pour.

Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il s'agit dans cet amendement de corriger une une iniquité. Entre étudiants en effet conformément à l'article. tirs 29 du code de l'éducation, les élèves admis au titre de l'aide au recrutement en classe préparatoire aux grandes écoles, des lycées de la défense sont tenus comme tous les étudiants d'ailleurs des classes préparatoires en grandes écoles, des lycées publics de s'inscrire parallèlement dans un établissement d'enseignement supérieur et cette inscription donne lieu au versement des droits d'inscription, prévue à l'article 719 tiré quatre du code de l'éducation, ainsi qu'au paiement de la contribution de vie étudiante et de Campus situé à l'article L. 841 du même code et donc les nous vous proposons de de corriger une iniquité existante entre étudiants en exonérant du paiement de cette contribution. Les élèves des lycées de défense qui viendraient à être exonérée des droits d'inscription dans le civil dans l'établissement d'enseignement supérieur sur des critères sociaux en effet les boursiers de l'enseignement supérieur sur critères sociaux sont actuellement exonérés de ces droits d'inscription et bénéficie que relativement d'une exonération de la contribution de vie étudiante du campus. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Avis favorable à un président. Monsieur le Ministre favorable je mets aux voix le 164 qui a reçu 2 avis favorable. Et pour. Qui compte. S'abstient il est adopté. Monsieur le Ministre, vous levez le gage. Il est levé. Article 18, le 256. Monsieur le Ministre. Oui, à un moment d'appel là aussi pour comprendre ce qui était décidé voté en commission. La double promotion fonctionnelle. Elle est prévue dans le texte pour les seuls officiers généraux, pour des raisons qu'on comprend bien qu'il tient aux particularités de la gestion du corps des officiers généraux là je vois qu'elle est étendue à l'ensemble. Des militaires. Et je ne vois pas quel besoin en matière de ressources humaines, cela correspond. Monsieur le rapporteur. Madame la présidente sur cet amendement, nous souhaitons donner un avis défavorable, parce que. Nos rapporteurs ont travaillé, notamment avec le Conseil supérieur de la fonction militaire et qui a évoqué, a plus de manière tout à fait formel, le fait que ce dispositif serait. Bénéfique pour des sous-officiers ou des officiers qui ne serait pas des officiers généraux et que l'on souhaiterait maintenir en en promotion. En double promotion fonctionnel en active donc proposer un avis défavorable. il est maintenu.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'aimerais vous faire changer d'avis sur cet amendement tend je le trouve frappée au coin du bon sens mais encore une fois je ne suis probablement pas objectif. Je vais essayer de vous donner avec un exemple relativement concret le le fait que ce soit assez intéressant de de de voter pour. En effet, dans la perspective d'un risque incendie d'un d'incendies accrus dans les territoires jusqu'alors épargnée par des incendies de forêt majeur qui était jusqu'alors cantonné plutôt sur la zone méditerranéenne et sur le Sud-Ouest. Cet amendement vise à identifier et à tester les pistes d'atterrissage pouvant permettre à des aéronefs de type Canadair Dash ou A400M qui peuvent désormais se charger en haut David taillés et de se ravitailler dans un périmètre restreint afin d'éteindre un incendie dans les meilleurs délais. C'est une sorte de rapprochement entre ce que pourrait faire la sécurité civile qui éviterait de construire de nouvelles infrastructures et en même temps ce serait gagnant pour nos nos armées qui avec des infrastructures militaires permettrait de les faire pérenniser. Je me permets de rappeler très rapidement les quantités d'eau un canadair c'est tonnes un Dash et 12 tonnes d'eau et un Kassem c'est 20, donc ça vaut quand même le coup de se poser la question et pour moi il y a pas de coûts engendrés. Pour le gouvernement, ni même pour les armées. Néanmoins, pour aboutir à une lutte efficace contre les incendies de forêt, il apparaît primordial de permettre à des moyens et reporté de bénéficier d'un maillage suffisamment dense de sites d'avitaillement. Pour cela, la présence de nombreuses pistes militaires ou tout du moins de nombreuses infrastructures militaires sur le territoire français est un atout qu'il s'agit de valoriser en y apportant aux abords, un dispositif d'avitaillement efficace permettant aux aéronefs de type Canadair d'âge ou à de se réapprovisionner en produit retardant la propagation de l'incendie. Le maintien en état des pistes et sous-jacent à cette utilisation par des appareils. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Avis de la commission. La commission a donné un avis favorable. Madame la présidente. Si Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. Oui. Or le le dialogue entre les 2 ministères Intérieur armées quand même satisfaisant sur. Cette affaire-là, est-ce que c'est la place de la LPM que d'écrire cela, moi je comprends la motivation sur le fond. Donc je m'en remets à la sagesse du Sénat pour être honnête. Pour être transparent sur le fond je que je je je je comprends ce que vous dites et j'en suis persuadé sur le fait qu'il fallait l'écrire dans la partie nord Mathilde loi de programmation militaire j'comme qui dirait un vieux d'août donc je m'en remets vraiment la sagesse du Sénat. Je vous laisse décider. Merci monsieur le ministre et je vais donc mettre aux voix l'amendement 171, rectifie qui a reçu un avis favorable de la commission. Sagesse du gouvernement qui. Pour. Qui compte. Qui s'abstient-il être adopté. Après l'article. Ah non. D'abord Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il est minuit je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demie afin de poursuivent l'examen de ce texte si vous en êtes d'accord et donc s'il y en a. Pas s'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé et nous continuons donc sur. Ce texte avec l'amendement 100. 72. Monsieur est toujours.

Cet amendement demande la rédaction par le gouvernement d'un rapport portant sur les capacités, une station des pistes implantées sur des zones militaires par des aéronefs dédié à la lutte contre les incendies de forêt ce rapport permettrait de déterminer également les besoins afin d'optimiser cet usage en cas de survenance d'incendies de forêt d'ampleur. Si Monsieur le. Ravi de la commission. Avis favorable madame. Favorable, Monsieur le Ministre. Sagesse renforcer. Une demande de rapport sur cette question utile mais hyper précise dans la partie nord massif de la LPM. Comme dirait le sénateur tu es mal qui a relu les anciennes LPM. Pour le coup de quelque chose de qui était quand même parti on peu bavard avec des grands objectifs stratégiques là on arrive à un degré de précision qui me paraît. Qui me très exigu une fois plus je dans la dynamique globale du texte. Depuis le début à l'Assemblée nationale. J'ai fait mon deuil d'avoir un, un texte nerveux et et un peu Sharper, donc allons-y sagesse. Alors je mets aux voix l'amendement 172 qui a reçu un avis favorable de la commission sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient il est adopté.

merci madame la présidente. Nos militaires passent régulièrement des examens libre médicaux et ils sont obligatoires pour entrer dans l'armée, mais ils sont également de mise avant de partir en mission à l'étranger par exemple.

Jusqu'ici tout va bien sauf que le médecin il faisait également mention de l'homosexualité de la Capitaine il écrivait ouvertement homosexuel, comme l'a révélé une enquête approfondie de France Info. Faire mention de l'orientation sexuelle sur la fiche n'ai rien d'autre qu'une stigmatisation afin d'éviter de tels cas dans le futur. Cet amendement du groupe écologiste et de ma collègue mais Mélanie Vogel, vise à interdire de mentionner l'orientation sexuelle dans le dossier individuel du militaire. La loi interdit déjà dimensionné des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à raison cet amendement compléterait cette liste pour éviter que de telles stigmatisations se reproduise au delà des fiches médicales cette interdiction s'appliquerait par ailleurs à tous les documents qui sont ajoutées aux dossiers individuels comme les décisions de congés ou les attestations émise après un exercice particulier. Cela me permet également de rappeler le rôle important que les médecins militaires peuvent jouer dans la lutte contre le harcèlement et le bizutage. On en parlait tout à l'heure dans l'armée. Ce sont ces médecins qui sont amenés à examiner les victimes et peuvent sonné la sonnette d'alarme et la plupart du temps il et elles le font et nous devons honorer leur travail infatigable merci. Monsieur le rapporteur. S'il vous plaît. Avis de la commission. Favorable à ma merci. Oui. Sagesse favorable. Alors je mets aux voix le 177 qui reçoit un avis favorable de la commission sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Ah. Le 20, amendement 121. Keffieh. C'est monsieur Cadic qui va le présenter. Merci madame la présidente. Dans le contexte de résurgence des tensions et compétitions internationales certains États étrangers étrangers n'hésitent pas à rechercher activement directement ou par l'intermédiaire d'entreprises agissant pour leur compte. La collaboration d'anciens militaires dont l'expertise technique ou le savoir-faire opérationnel présente un intérêt stratégique pour le développement de leurs propres capacités militaires. L'article 20 vise à instituer un contrôle préventif et dissuasif concernant les militaires ou anciens militaires ayant occupé des fonctions d'une sensibilité particulière et souhaitant exercer une activité lucrative pour le compte d'un État étranger ou d'une entreprise étrangère ou sous contrôle étranger. Intervenant dans le domaine de la défense et de la sécurité. Le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux diplomates ayant le grade de ministre plénipotentiaire. Je fais souvent. L'analogie entre la justice. Et l'intérieur. Eh bien la diplomatie. Les affaires étrangères sont à la Défense. La même chose. Et les diplomates. Les ambassadeurs ont un rôle. Éminent. Et lorsque eux-mêmes un sorte du service et se mettent à la disposition d'une, d'un service d'un pays étranger, hé bien l'impact peut être aussi dommageable qu'avec des militaires et c'est le sens de cet amendement, je vous remercie. Merci cher collègue. Monsieur le rapporteur. Avis de la commission. l'amendement porte sur les diplomates ayant le grade de ministre ni potentiel. Or, je crois me souvenir que le corps des ministe plénipotentiaire a été supprimée par le gouvernement dans le cadre de la réforme du corps diplomatique. Monsieur le ministre. Merci beaucoup madame la présidente. De fait, ça pose la question de la de l'amendement, c'est. Tous les. Autres corps de métier. Qui pourrait avoir accès à un savoir faire militaire. Bon. Comme je l'ai indiqué plusieurs fois à l'Assemblée. Déjà le seul fait qu'on introduise dans le droit. Ces mesures sont déjà stupéfiante parce que ça n'a jamais, jamais été fait auparavant hein. Je vous rappelle que la c'est c'est le au fond pour traiter les sujets de pilotes initialement puis on est allé au-delà et dans l'assemblée, enfin dans le débat à l'Assemblée. Pardonnez-moi, on a évidemment durcit la mesure. Donc, au-delà du fait que cette affaire de ministre. Puis une potentielle enfin. En quoi le grade de ministre et plénipotentiaire d'ailleurs vous donne accès à un savoir faire militaire particulier. Vous avez d'autres diplomates dans un poste diplomatique qui ne sont pas Ministre plénipotentiaire et qui peuvent travailler en lien avec la mission de défense ou avec la cellule. Le cas échéant, le poste de DGSE du coin. Donc en fait le grade de ministre plénipotentiaire en tant que telle.

Y compris d'ailleurs si on on va là aussi. Pour certains emplois. Dans d'autres administrations que le ministère des Armées. La réflexion méritera d'être posé. Et au fond, on voit bien quand même que cette loi de programmation militaire elle pose un 1er parpaing mais je suis sûr que ceux qui nous succéderont ils reviendront sur sur d'autres thématiques. Voilà donc en l'espèce parce que l'amendement été hyper précis. Je pense qu'il faut faire défavorable aux demandes de retrait mais cela n'interdit pas la réflexion à l'avenir. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur K. Dick. Monsieur le Ministre, effectivement les diplomates. Et vous le savez peuvent contribuer à l'influence. Et la guerre d'influence. Est aussi aujourd'hui palpable que le conflit telle qu'on le fait le le voit sur les théâtres d'opérations. J'entends noté effectivement par rapport à ce qui a été dit ce matin de la part de la commission que il y a eu un travail et donc un regard qui peut différent donc évidemment je vais le retirer, mais simplement il me semble vraiment important qu'on prenne en compte cette dimension parce que pour assister à un certain nombre de conférences. Quand je vois effectivement des diplomates qui servait la France et qui se mettent à reprendre le verbatim de puissances étrangères qui ne ne veulent pas que du bien, ça me gêne. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, je vous remercie. Si cher collègue, et donc l'amendement 121 rectifié et retiré. Nous passons à l'examen de l'amendement 257 du gouvernement, Monsieur le Ministre.

Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Donc l'initiative de notre collègue. Jérôme Bascher. Et plusieurs. D'entre nous concernant cet amendement. Il fait référence à la délégation parlementaire au rang renseignements qui est, qui En octobre 2007, l'émission de cette délégation parlementaire anciennement ne couvre pas le renseignement économique c'est aussi une lacune dans le contrôle démocratique qui doit être. Comblé.

pour faire entendre des personnalités compétentes sur des sujets différents. Sur ces différents sujets et adresser des recommandations et observations au président de la République au 1er ministre ainsi qu'aux ministres afin de préserver les compétences d'autres organes au Parlement du Parlement. Il a précisé que cette délégation exercerait ses compétences sous réserve de celle de la délégation parlementaire au renseignement. Quel est l'objet de cet amendement. pardon pardon pardon, pardon monsieur le rapporteur. Je fais une bêtise. Nous sommes en discussion commune et donc il y a encore l'amendement de madame Gréaume a présenté. Merci. Dans un objectif de transparence, il nous sommes tout à fait sain dans une démocratie, que le gouvernement doivent rendre des comptes sur des politiques ayant des impacts sur les intérêts économiques. Scientifique de la nation en comme ici à en commission l'idée de la création d'une telle délégation fut balayé au motif que celle-ci empiéteraient sur la délégation parlementaire au renseignement voire même risquerait d'émietter le contrôle parlementaire en matière de renseignement opposé ainsi l'existence de la délégation au renseignement et celle de la à la sécurité économique relève selon moi d'un non-sens en effet la délégation au renseignement du dispose de prérogatives pour traiter de questions économiques toutefois le Champ de compétence de cette délégation étant large, très large. Cela conduit à ne pas traiter en profondeur les sujets économiques. Et puis une délégation à la sécurité économique et aux investissements ne disposait pas d'un pouvoir de contrôle sur le gouvernement de même nature que celle sur le renseignement, l'une exerce. Un contrôle a priori, tandis que la seconde exercerait un contrôle a posteriori l'idée de créer une telle délégation c'est justement de se prémunir contre toute atteinte à des secteurs. Qu'au courant à la souveraineté de la France et non de les constater une fois que le mal soit fait par exemple sur le sujet du numérique comme nous avons pu le montrer à travers quelques-uns de nos amendements. Le numérique constitue un secteur stratégique tant pour notre industrie militaire que pour celle du civil et plus généralement pour l'ensemble de nos institutions publiques s'atteler à ce que l'État investisse dans ce secteur reconstruisent les filières industrielles régalienne du secteur et ici je pense notamment à STMicro SoiTec et cetera nécessite à la fois de l'arrêt de la réactivité, mais aussi la participation de la représentation nationale la question industrielle et la question de la souveraineté nécessitent une large mobilisation du pays et celle-ci doit s'exprimer par la voix de ses parlementaires merci. Merci madame Gréaume. Hein, voilà maintenant monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Non, faire une réponse commune pour ces deux amendements. La création d'une délégation parlementaire à la sécurité économique empiéteraient manifestement sur les compétences de plusieurs commissions permanentes et sur celle de la délégation parlementaire au renseignement qui du reste a déjà produit, je crois me souvenir sous la présidence de Philippe Bas. Un rapport tout à fait passionnant sur les sujets d'ingérence économique de captation des secrets industriels et donc que tout ceci entrent dans le Champ de la délégation parlementaire au renseignement. au renseignement. C'est donc un avis défavorable aux deux amendements. Monsieur le ministre un avis du gouvernement. Oui des défavorable. Même si. Pour la forme, je préfère taire sagesse. Dans la mesure où comme il s'agit d'organisation interne au Parlement. On nous la séparation du pouvoir. J'estime heureux que le gouvernement ne donne pas des vitraux définitif. J'ai fait la même chose à l'Assemblée sur des problèmes entre la commission des affaires étrangères et la Commission de la Défense. Moi en tout cas je me range. À titre personnel, je me range à l'avis du rapporteur, président. Merci monsieur le ministre. Monsieur le président du fait, a demandé la parole pour explication de vote. Volontiers, même la présidente simplement pour donner la commission des Lois s'est saisie pour avis. De cette demande. C'est évidemment un avis extrêmement défavorable. La délégation parlementaire au renseignement fait rempli cette mission en 2018, elle a rendu un 1er rapport gageons que peut-être dans les semaines, les mois qui viennent il y aura d'autres rapports de cette nature. Elle bénéficie du lieu du liée au secret de la défense qui est absolument essentiel également aux moyens techniques a tous les moyens qui lui permettent d'avoir à connaître cette situation, dans ces conditions là il est inutile de créer des délégations supplémentaires qui sont de nature d'ailleurs à disperser. Y compris le la maîtrise de l'information et la qualité des relations qui existent à la fois que les services de renseignement et avec le gouvernement. Donc, la commission des lois a émis un avis très défavorable à cet amendement. Si monsieur le président, monsieur.

Compétent du à la fois de Monsieur le Ministre des et, des 2 présidents de commissions, commission, Défense, Affaires étrangères et commissions des lois je le retire. La mini-donc le 60. Effectif. S'il est retiré. Monsieur le président Laurent vous souhaitiez prendre la parole pour explication de vote. Oui, ce que dit le président. Quand mon des des n'est pas fausse. C'est c'est à cheval sur des compétences qui existe dans des. Dans des commissions permanentes actuel mais le problème c'est que il nous manque parfois justement un regard transversal sur ces questions. Et que. Le regard qui peut être celui de la commission des affaires économiques ou celui de la Direction du renseignement dans le domaine militaire ne croissent pas suffisamment. Les choses pour s'apercevoir que un problème de sécurité économique touchant à notre souveraineté est en train de se faire jour et de prendre des proportions qui peuvent être très importantes. Donc ah regard stratégique transversal que permettrait cette délégation serait à nos yeux, extrêmement utile. Donc nous maintenons l'amendement. Si cher collègue, et donc je vais mettre aux voix l'amendement 151 rectifié qui a reçu un avis défavorable de la commission et sagesse défavorable du tout j'ai cru comprendre du gouvernement. Très bien. Monsieur le Ministre, je n'ai rien dit, c'est vous qui le dites. Et donc qu'il est. Qui est contre. Il s'abstient. Il n'est pas adopté, je me vois l'article 22 quater qui et pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Article. Le 22 quater amendement 258 du gouvernement, Monsieur le Ministre défendu. Défendu monsieur le rapporteur. Ça aurait pu donner lieu à un long débat. C'est un amendement qui résulte de de la mise en application des recommandations de la CNCTR qui avaient été formulées dans son rapport public de juin 2023, c'est-à-dire il y a quelques semaines. le gouvernement propose. De supprimer le contrôle permanent et immédiat de la CNCTR sur les données conservées par les services. La position de la Commission est sensiblement différente, puisqu'elle a introduit le droit pour la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement d'accéder à distance et de manière permanente aux données conservées par les services de renseignement sans avoir à se déplacer. Un long débat sur lequel. La commission s'est exprimé, amendement un avis défavorable à l'amendement du gouvernement. Merci monsieur le rapporteur. Explications de vote de Monsieur le Président buffet. Oui madame la présidente. Sur ce point, je pense que ça mérite des précisions. Elle avait évoqué à l'occasion de la discussion générale. En début d'après-midi. Quel est le sujet les services utilisent de plus en plus de moyens intrusifs pour avoir les renseignements qui leur sont utiles pour mener leur action. Il n'est pas question évidemment de remettre en cause ces moyens. Les moyens traditionnels sont contrôlés par. Ce qu'on appelle le l'organisme logique à circonstance là, ils ne sont pas sur ses moyens les plus intrusif pour des questions d'adaptation. L'idée, c'est de permettre à la CNCTR de d'assurer ce contrôle. Elle le fait habituellement auprès du GIC pourrait tout à fait clair. Il faut donc lui permettre aussi de contrôler ses moyens les plus intrusif. Une fois de plus, c'est pas pour remettre en cause les capacités à agir, elles sont nécessaires et on a besoin de ce contrôle. Bon, la question qui se pose, monsieur le ministre, on a compris. C'est la question de la mise en oeuvre, c'est moi la question du principe que de la question de la mise en oeuvre dans ces cas-là, trouvons un délai. Déterminé un délai communément on l'inscrit dans le texte et de ce fait, on n'aura pas de difficulté des discussions qui émane des auditions que nous avons eu une fois de plus, je le redis, dans pas en cause le principe mais le délai de mise en oeuvre qui. Dont on peut bien comprendre est compliqué à faire long. Mais il ne faut pas se priver de le faire, il faut avancer un peu, faut avancer sur ce dossier. Je crois que c'est pour la sécurité, tout le monde des services. Bien évidemment mais aussi chacun de concitoyens. Si Monsieur le Président. S'il n'y a plus de demandes d'explications de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 258 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il n'est pas adopté, je me vois l'article 22 quater qui et pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Article 23 amendement du gouvernement numéro 259. Défendu à la présidente. Oui monsieur le rapporteur favorable je mets aux voix cet amendement donc avec un avis favorable qui pour qui compte qui s'abstient il est adopté le 153 présenté par monsieur Laurent. Oui, l'article 23 entreprend une réécriture complète du régime des réquisitions. Celui-ci est activable en cas de menace actuelle ou prévisible et la notion de menace prévisible nous semble tout de même beaucoup plus flou. De la même manière, la liste des motifs d'activation du régime est relativement longue et peut couvrir des situations extrêmement diverses. Or les réquisitions, rappelant rappelons-le empiète tout de même lourdement sur les libertés aussi nous semble important. D'assortir ce nouveau régime des réquisitions d'une sécurité démocratique supplémentaire. En prévoyant pour les réquisitions entreprises sur le fondement d'une menace prévisible une validation par le Parlement. C'est le sens de cet amendement.

l'article 23 nous paraît équilibré. Elle donne en effet au juge les moyens de contrôler la la pertinence des mesures de réquisition au regard des objectifs poursuivis et des circonstances de temps et de lieu. Je rappelle ce dispositif. Le Parlement se prononce sur le régime des réquisitions sur la base de l'article 23 l'exécutif met en oeuvre ses réquisitions, le juge contrôle les mesures prises chacun des trois pouvoirs est dans son rôle et le Parlement dispose de pouvoirs de contrôle sur l'action de l'exécutif, avis défavorable.

qui compte qui s'abstient il est adopté. Après l'article 23. Nous avons. 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 112 madame Duranton. Merci madame la présidente, là encore, il s'agit de faire évoluer les dispositions existantes pour retrouver de l'agilité et de la fluidité dans le cadre d'une compétition internationale en matière de normes, il est primordial d'avoir des institutions réactive qui protégeront notre savoir-faire et les droits de la propriété, indique-t-elle actuelle des déposants. Donc cet amendement vise donc à transférer la compétence résiduelle du ministre chargé de la propriété industrielle au directeur de l'Institut national de la propriété intellectuelle, comme c'est déjà le cas pour les brevets nationaux afin d'économiser du temps et des dépenses que nos entreprises pourront réaffecter plus utilement. Merci madame la présidente, monsieur Ministre amendements identiques. Mais merci. Pas tout à fait, mais même explication. Heure monsieur le. Rapporteur avis de la commission sur ces 2. La Commission sollicite l'avis du gouvernement sur ces deux amendements. Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. Hé bien, avis favorable au 112. Et demande de retrait du 176 au bénéfice du 112 pour des raisons purement rédactionnelles dispositif.

j'ai pas demandé. Monsieur le rapporteur. Vous ranger à l'avis de Monsieur le Ministre donc je mets aux voix l'amendement 112 qui reçoit un avis favorable. De la commission. Et du gouvernement. Qui est pour.

Voilà. Et donc, article 24. 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 298. Monsieur Cambon monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. Cet amendement a pour objet d'inclure la notion de consultation de l'entreprise concernée dans les dispositifs prévus aux articles 1339 1 et 2 du code de la défense qui ont été créés par ce projet de loi afin d'assurer la prise en compte des impératifs et des suggestions s'imposant par ailleurs à la dite entreprise. C'est une demande très soutenue de la part de nos entreprises de défense en la matière. Merci monsieur le rapporteur. Il me semble que le 184 rectifié n'ait pas défendu il tomba. Le 260. Monsieur le Ministre, amendement du gouvernement. Oui alors il est défendu. On est dans une discussion commune mais quand même pas tous complètement la même chose pour être honnête On y reviendra pour les avions. Cet amendement précise les modalités d'application du principe de proportionnalité au mécanisme de constitution des stocks stratégiques, il modifie l'actuelle rédaction de l'article 24. Qui prévoyait que la valeur du stock prescrit ne pouvait pas excéder une proportion maximale du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc cet amendement prévoit en août une prise en compte de la situation économique des entreprises soumises à l'obligation de ces constitution de stocks stratégiques. Il prévoit aussi que le volume des stocks ne peut excéder une durée maximale de 24 mois de couverture des besoins d'approvisionnements et d'une manière générale, la prise en compte des conditions générales d'approvisionnement et de conservation de la matière du composant du rechange et du produits semi-finis ces précisions sont de nature à renforcer les garanties apportées aux entreprises qui vont être concernés par l'obligation de constituer des stocks. Et voilà donc cet amendement de 199. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Peut être nous donner tout de suite l'avis de la commission sur le 260. C'est un amendement qui est légèrement différent de l'amendement 299 donc je préférerais évidemment l'amendement 299 et je donne un avis défavorable à celui-ci de aux 260. Merci monsieur le rapporteur. Et Monsieur le Ministre, donc la vie sur les deux amendements de la commission. Alors. Sur le 298 et sur le 184.000 n'même pas été défendue. Pour le coup, pour moi il est déjà satisfait donc avis défavorable je. Ne vois pas ce que ça apporte en tant que telle et après quand on la rédaction. Son je sais quand on a mon nom vient du gouvernement, il a peu de chances d'aboutir. Donc je le maintiens quand même. C'est le défenseur avec sa femme. Très bien alors je mets tout d'abord aux voix l'amendement 298. De la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

en fait nous sommes défavorables à cet amendement parce que les munitions qui constituent les produits finis ne peuvent pas rentrer dans la liste des stocks pouvant être constitué. Je propose de retirer cet amendement sinon nous serons des favoris.

je vous propose qu'on termine l'article. Si tout et ça rapidement, il nous reste. Trois amendements, si vous le voulez bien. Merci madame présente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais être très rapide. Cet amendement vise à encourager l'autorité administrative a sollicité les entreprises françaises ou a minima européenne afin d'approvisionner son stock de munitions de matière ou composants d'intérêt stratégique. Si je peux me de un et un exemple par exemple aujourd'hui sur de la petite munition on achète essentiellement Israël avec des munitions fabriquées par des machines françaises en passant par la Belgique. Donc aujourd'hui. Avoir des machines de munitions fabriquées en France et pouvoir développer l'industrie missionnaire en France serait une très bonne chose donc privilégier les entreprises de notre base industrielle et technologique constituera une première étape vers la constitution d'une industrie munitions nerfs française clairement identifiés, étape indispensable vers une forme de souveraineté dans l'industrie munis scionner. Si avis de la commission. Pour les mêmes raisons que l'amendement précédent la veille et défavorable puisque les munitions, c'est un produit fini. Le ministre défavorable et ma vie. Je mets aux voix le 169 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il n'est pas adopté le 261. Il était. Entendu, monsieur le rapporteur. Avis de la commission sur l'amendement du. Un avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement 261 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour.

D'instaurer une consultation obligatoire et systématique du président de la Polynésie française par le ministère des Armées. Dès lors que les ressources naturelles de la Polynésie sont en jeu. Quand bien même ses ressources devait être devrait devrait être qualifié de matières premières stratégiques actuellement l'article 14 du statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que l'État est seul compétent. S'agissant des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République. Or la détermination des dites matières premières stratégiques relève exclusivement de l'état qui est libre y inclure par exemple les éléments de Terres rares dont les fonds marins polynésiens sont particulièrement riche. Pourtant, selon l'article 47 de ce même statut d'autonomie. Il appartient à la Polynésie française d'exercer de réglementer l'exploitation de ces ressources naturelles biologique et non biologique, notamment celle du sol et du sous-sol de sa zone économique exclusive. De même, par des résolutions annuel de son assemblée générale depuis 2013, l'ONU ne cesse d'exhorter la France. À garantir la souveraineté permanente du peuple polynésien à l'égard des ses ressources naturelles comprenant ces ressources marines et sous-marine. Et donc l'ensemble des Terres rares qui s'y trouvent. C'est donc le sens de notre amendement. Si Monsieur le Président et maintenant l'avis de la commission sur cet amendement. Alors c'est une demande de retrait ou un avis défavorable d'abord parce qu'on se demande pourquoi cet amendement vise à circonscrire une cette obligation à la seule Polynésie française par ailleurs s'agissant de matières premières stratégiques il nous sommes très important de limiter le plus possible notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, avis défavorable aussi non retrait. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. Oui. Avis défavorable je quand j'entends peuple polynésien. Comment avec nos concitoyens polynésien ne font partie que d'un seul peuple au peuple français. Je vous remercie et je mets aux voix l'amendement 154 qui a reçu 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je mets aux voix. L'article 24 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Monsieur Cigolotti vous avez la parole. Vous me permettrez j'espère une petite digression à nos débats et je voulais, au nom du groupe Union centriste. Saluer notre président une autre collègue Valérie Létard dont c'était ce soir la dernière présidence de séance et l'a remercié pour son investissement.

Eh bien, chers collègues, j'avais donc levé la séance. Nous avons examiné 94 amendements cours de la journée. Il en reste 192 examiner sur ce texte. Prochaine séance mercredi 28 juin à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.